La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 15 avril 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. j'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Henri Goetschy, qui fut sénateur du Haut-Rhin de 1977 à 1995, et Marc Bécam,

Cette initiative, conjointe avec nos collègues Les Républicains de l'Assemblée nationale, se veut constructive, dans un contexte économique et social qui ne permet pas de faux pas et exige de clarifier le débat public. Avant même d'entrer dans le détail de ce sujet, je souhaiterais que nous fassions l'effort collectif de toujours nous interroger sur la motivation et l'opportunité de toute modification de la loi. L'instabilité législative que nous portons potentiellement, à chaque texte, est-elle justifiée par l'intérêt général ? Dans le cas qui nous intéresse, est-il opportun de porter une réforme susceptible de déstabiliser un élément fondateur de la protection des salariés et des entreprises ? Alors que nous sommes « face au mur des faillites », pour reprendre l'expression d'une étude récemment publiée, comment justifier de risquer de remettre en cause la pérennité de l'AGS ? Pourquoi prendre un tel risque, alors que la destruction de 750 000 emplois est évoquée et que les projections sont pessimistes ? Le cabinet Euler Hermes prévoit une hausse de 32 % des défaillances d'entreprise en 2021, tandis que Coface estime que 22 000 entreprises ont survécu uniquement grâce aux aides et devraient mettre la clé sous la porte d'ici à 2022.

Ne se contentant pas de limiter le texte aux ajustements nécessaires pour clarifier le droit et le coordonner aux évolutions européennes, le Gouvernement a ainsi voulu proposer un nouvel agencement de l'article L. 643-8 du code de commerce, débouchant sur ce que de nombreux commentateurs ont qualifié de « rétrogradation » de la créance superprivilégiée de l'AGS. Je rappelle que les procédures collectives font en effet intervenir plusieurs acteurs, sous l'autorité du tribunal de commerce. Outre l'entreprise, il s'agit des administrateurs et mandataires judiciaires, des autres praticiens de la procédure et des créanciers de l'entreprise, qu'ils soient publics ou privés. L'actuel régime de garantie des salaires, créé en 1973 à l'initiative des employeurs qui le financent, est le principal créancier institutionnel privé. L'AGS assure, en vertu de la loi, l'avance des créances salariales, à savoir les salaires antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais aussi les indemnités de licenciement, de préavis ou de congés payés. L'AGS engage ensuite, dans le cadre de la procédure collective, un processus de récupération des sommes avancées, avec un superprivilège prévu par la loi. Le régime de garantie des salaires en France est un élément essentiel de notre droit des entreprises en difficulté, avec un objectif en termes d'emplois.

qui permet de préserver l'emploi et de maintenir la viabilité économique des entreprises en difficulté, mais aussi, plus largement, de soutenir le rebond de l'activité économique française. Pour résumer le nouvel ordre proposé par le projet d'ordonnance pour les créances,

ces frais sont critiqués pour leur niveau parfois excessif, leur manque de transparence et de contrôle. En effet, les abus de certains, dans quelques procédures, ne cessent de jeter l'opprobre sur l'ensemble de ces professionnels. L'absence de contrôle laisse régulièrement la place libre à des situations maintes fois dénoncées, depuis Arnaud Montebourg en 2001 jusqu'à Richard Ferrand plus récemment, ou encore l'Autorité de la concurrence. Dans un contexte de crise économique sans précédent, comment pourrions-nous ne pas être choqués par un tel projet d'ordonnance, d'autant que la réforme proposée par la Chancellerie, en rétrogradant la place des créances de l'AGS, remettrait en cause sa pérennité économique Les projections de récupération des créances ainsi déclassées situent la perte à 300 millions ou 400 millions d'euros par an. Par conséquent, seules deux options seraient alors possibles. La première serait de réduire le périmètre de prise en charge par l'AGS, en amputant les sommes perçues ou en excluant certaines dépenses. serait de relever substantiellement le taux de cotisation des entreprises en le triplant. Aucune de ces hypothèses ne nous paraît acceptable dans cette période de crise, où de très nombreuses entreprises, notamment les TPE et PME, luttent pour survivre.

Pourquoi vouloir prendre le risque d'un tel bouleversement en pleine crise économique ? Où est l'intérêt général dans cette démarche ? Vous avez fort heureusement confié une mission à René Ricol, qui a su réintroduire du bon sens et évoquer des chantiers pour l'avenir. La « sagesse » sénatoriale salue celle de M. Ricol, qui demande le maintien à droit constant du privilège dont bénéficie aujourd'hui l'AGS. Il est urgent de ne rien changer pour garantir la pérennité de notre système, l'un des plus protecteurs de l'emploi en Europe. Les réformes non imposées par la transposition de la directive doivent être appréhendées dans le cadre d'un projet de loi, et non subrepticement par le biais d'une ordonnance. Le Sénat sera heureux de s'y associer, en prenant notamment en compte les travaux de nos collègues de la commission des lois sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, qui seront présentés le 19 mai prochain. Comme le souligne M. Ricol, et ainsi que nous l'avions fait dans notre proposition de résolution, il est essentiel aujourd'hui d'élargir le débat à d'autres sujets, alors que tout le monde s'attend à des défaillances d'entreprise en cascade. Ainsi, pourquoi ne pas envisager un rôle élargi de l'AGS dans les mesures de reclassement des salariés ou dans les procédures de prévention ? Pourquoi ne pas prévoir son intervention auprès des groupements d'employeurs- aujourd'hui d'amortisseur social pour leurs membres en difficulté, mais ils ont rarement la solidité financière pour assumer ce rôle en cas de difficultés à la chaîne Et pourquoi ne pas faire intervenir l'AGS pour garantir les sommes dues aux travailleurs indépendants, trop souvent exclus des mesures visant à soutenir l'emploi ? D'autres sujets nous semblent également prioritaires compte tenu de la situation de crise que traversent nos entreprises, notamment les TPE et PME. Pourquoi ne pas créer une fois pour toutes les conditions de la transparence et d'un contrôle raisonnable des frais de l'ensemble des professionnels intervenant dans les procédures collectives ? N'est-il pas urgent de définir un cadre permettant de faire évoluer les pratiques ? Enfin, compte tenu des délais observés pour mener à bien certaines procédures collectives, pourquoi ne pas prévoir des formules simplifiées et accélérées, notre délégation aux entreprises le préconisait déjà, il y a trois ans, dans un rapport de notre collègue Olivier Cadic sur la liberté d'entreprendre ? Madame la ministre, le groupe Les Républicains espère que vous pourrez, bien

Les enjeux sont trop importants pour que nous puissions nous en accommoder. Mes chers collègues, compte tenu de la gravité de la situation économique et sociale, je vous demande de voter en faveur de la proposition de résolution n° 463

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons à présent concerne l'avenir d'un mécanisme éprouvé et essentiel pour le monde économique : le régime de garantie des salaires. Nous avons la chance de disposer en France d'un système parmi les plus protecteurs en Europe, permettant de garantir le versement des salaires lorsqu'une entreprise placée en procédure collective n'est plus en mesure de le faire. L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est approvisionnée par un double financement : les cotisations patronales, d'une part ; les créances prises sur les entreprises, d'autre part. Ce dernier financement, représentant 36 % de ses ressources en 2019, est possible grâce au superprivilège dont bénéficie l'AGS, qui lui permet de figurer au troisième rang dans l'ordre des créanciers. Cette pratique est actuellement remise en question du fait d'un conflit ouvert entre le régime de garantie des salaires et les administrateurs et mandataires judiciaires. Jusqu'à présent, l'AGS s'engageait à restituer sur demande les fonds nécessaires à la couverture des frais de justice et de procédure. À la suite d'abus constatés, l'AGS refuse désormais de payer ces avances. Le projet de réforme préparé par le ministère de la justice prévoit de transposer la directive européenne Restructuration et insolvabilité, adoptée le 20 juin 2019. Elle introduirait des classes de créanciers et conduirait à rétrograder le rang de l'AGS dans l'ordre des créanciers à la sixième position, au profit des administrateurs et mandataires judiciaires qui en ont fait la demande. Cette réforme, si elle était adoptée en l'état, fragiliserait le financement de la garantie des salaires et conduirait à une hausse du taux des cotisations patronales ou à une réduction de la prise en charge des salaires. Ce déséquilibre financier à venir est d'autant plus dommageable qu'il intervient en pleine crise sanitaire, laquelle entraîne non seulement une diminution de 9 % des comptes de l'AGS, du fait des mesures de chômage partiel, mais fragilise aussi l'ensemble du monde économique. Le mois de mars dernier a été marqué par une explosion du nombre de liquidations directes d'entreprises en cessation de paiements, avec une hausse de 155 % des défaillances.

Les effets de la pandémie sur les économies vont se répercuter à long terme. La BCE anticipe une vague d'insolvabilités et préconise de cibler les aides publiques sur les entreprises viables, susceptibles de survivre sans le soutien des États. Avec la fin des aides et le retour à la normale de l'activité économique, la France pourrait comptabiliser 22 000 entreprises non viables. Aussi est-il plus que jamais indispensable de conserver le système de garantie AGS, institué par la loi du 27 décembre 1973. Cette procédure joue depuis des années un rôle d'amortisseur social et contribue au financement des entreprises en faillite. Le récent rapport sur le sujet remis par René Ricol au Gouvernement va dans le sens d'une préservation de la priorité du paiement des salaires sur le financement des honoraires des administrateurs et mandataires judiciaires. L'AGS garantit chaque année le versement de leur salaire à plus de 150 000 salariés. L'avant-projet de réforme dégraderait directement la situation financière des salariés concernés par des faillites. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il doit évoluer afin de préserver le superprivilège des salariés en cas de liquidation judiciaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution de notre collègue prolonge le rapport de René Ricol remis au Premier ministre à la suite des premières réactions sur le projet d'ordonnance du ministère de la justice justice visant à transposer la directive européenne Restructuration et insolvabilité, sur fond de dégradation des relations entre les administrateurs et mandataires judiciaires et l'AGS. Le rapport Ricol confirme qu'une mesure de ce projet, largement contestée par les organisations syndicales des salariés et du patronat, rétrograderait l'AGS derrière les frais de justice en cas de liquidation judiciaire. Le projet d'ordonnance ne se ferait dès lors plus à droit constant, avec des créances salariales superprivilégiées, puis le paiement des frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture. Rien n'oblige pourtant le projet de transposition à modifier l'ordre des créanciers privilégiés, la directive européenne ne comprenant pas d'objectif d'harmonisation de résolution vise, au contraire, à maintenir l'état actuel du droit. Le groupe écologiste soutient cette position, soucieux de défendre un outil efficace de protection de salariés déjà éprouvés lors des procédures collectives.

pourrait aussi être requis pour rétablir l'équilibre, ce qui inquiète l'organisation patronale. Le taux de couverture des avances de créances salariales par les recettes de cotisations patronales nettement baissé depuis 2017. Ajouté aux récupérations, il assure à peine l'équilibre du régime. La modification de l'ordre des créances ferait ainsi définitivement basculer le régime dans le déséquilibre financier.

La trésorerie du régime sera touchée, ce qui rendra difficile le maintien de la réactivité de paiement aux mandataires, et donc aux salariés, caractéristique du régime français. la crise sociale actuelle et à venir ne saurait être aggravée par l'affaiblissement du rôle d'amortisseur social de l'AGS au sein de notre protection sociale. Le maintien des créances

d'oeuvrer à plus de transparence, de maîtrise et de contrôle des frais de justice. Tous les acteurs des procédures collectives se disent néanmoins attachés à la pérennité de notre système de garantie. Nous devons donc parvenir

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte déposé par M. le président Bruno Retailleau et plusieurs membres du groupe Les Républicains témoigne de la préoccupation que les parlementaires peuvent avoir pour les entreprises et salariés de notre pays. ce projet d'ordonnance pourrait mettre en péril le paiement des salariés dont les entreprises seraient en situation de faillite. Vous n'êtes pas les seuls à avoir pointé cette limite, mes chers collègues. Dans un climat à haut risque de faillite, votre préoccupation est parfaitement justifiée.

me semble ensuite essentiel de mettre en lumière le travail de concertation, pour s'assurer que toutes les parties prenantes participent à la rédaction des ordonnances, notamment au vu des répercussions que celles-ci pourront pourront avoir. L'AGS, en 2019, c'est 1,5 milliard d'euros avancés, 182 000 salariés bénéficiaires, la quasi-totalité des avances versées dans un délai de cinq jours et un régime de protection des créances des salariés qui ne coûte pas un centime au contribuable. un centime au contribuable. Cela a été rappelé, l'efficacité de ce système de garantie des salaires tient pour partie au superprivilège dont jouit l'AGS. Celle-ci apparaît comme prioritaire dans l'ordre des créanciers d'une entreprise en procédure collective, bien que cet ordre ne soit pas explicitement établi. C'est d'ailleurs l'intégration d'un ordre explicite qui est à la source de la difficulté, car les pratiques existantes ne sont pas clairement définies par un cadre réglementé. Une telle déstabilisation du régime de garantie des salaires pourrait conduire à l'ébranlement de l'équilibre financier de l'AGS, et donc avoir des répercussions sur son rôle envers les salariés d'entreprises en faillite. Pour autant, notons que les paiements à l'échéance des frais judiciaires précèdent déjà les récupérations au profit

M. Ricol l'exprime clairement dans son rapport : « [Si] la protection des créances salariales constitue un enjeu majeur dans le dispositif français, l'efficacité des procédures collectives doit aussi être un objectif essentiel. » Cet équilibre, nécessaire, doit être protégé. Oui, la rétrogradation à un rang inférieur dans l'ordre des créanciers pourrait avoir comme effet de réduire mécaniquement les remboursements de créances que l'AGS parvient à récupérer. Aussi, le Premier ministre a confié à René Ricol une mission sur l'articulation entre le régime de garantie des salaires et le rôle des administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures collectives. Le rapport, rendu le 15 avril dernier, traite tout particulièrement de l'implication pour l'AGS de la transposition de la directive européenne et présente des recommandations pour améliorer l'avant-projet d'ordonnance.

Il est donc nécessaire de s'appuyer sur les conclusions du rapport Ricol, qui suggère un compromis consistant à écouter les craintes des partenaires sociaux tout en permettant une transposition adéquate de la directive. Ce projet d'ordonnance permettra de clarifier les interprétations aujourd'hui divergentes du droit sur l'articulation entre les frais de justice et les remboursements de l'AGS, au bénéfice d'une meilleure lisibilité pour toutes les parties prenantes.

Pour autant, je comprends votre souhait de soumettre aujourd'hui ce texte à notre vote, mes chers collègues. Les résolutions constituent sans nul doute l'une des voies d'affirmation du Parlement, en permettant une expression distincte de la réponse législative.

le Premier ministre, « l'AGS est un élément essentiel de l'organisation des procédures françaises, auquel le Gouvernement est très attaché ». Le rôle essentiel de notre système de garantie des salaires étant ainsi réaffirmé,

La prolongation du fonds de solidarité mis en place pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et par les mesures de confinement jusqu'au 30 juin 2021 en est un exemple.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'AGS, dont nous discutons aujourd'hui, est une structure qui, bien qu'imparfaite dans sa gestion, est fondamentale pour les salariés et les entreprises. Pourtant, elle est aujourd'hui menacée par une réforme à laquelle s'opposent des organisations syndicales et patronales. Je remercie sincèrement nos collègues Bruno Retailleau et Serge Babary, ainsi que l'ensemble du groupe Les Républicains, de nous donner l'occasion d'affirmer ici la nécessité de préserver cette association essentielle. Créée en 1973, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dite AGS, garantit le versement de leurs salaires aux employés d'une entreprise en liquidation judiciaire, si celle-ci ne peut les prendre en charge. Rien qu'en 2019, 1,5 milliard d'euros ont été avancés à 182 000 salariés et la quasi-totalité des avances a été versée dans un délai de cinq jours. En ces temps de crise sanitaire, sociale et économique, dont les effets se feront sentir de manière durable, l'utilité de ce régime et son caractère fondamental ne peuvent être remis en cause. L'AGS a été créée pour protéger les salariés, non pour payer les frais de justice : il est donc important de lui conserver son but initial, d'autant que, dans cette crise comme dans toutes les autres, les salariés se trouvent en première ligne. En outre, on ne compte plus les licenciements survenus au cours des derniers mois. Mais surtout, c'est un second coup dur pour le monde salarial, car à la casse programmée du modèle de l'AGS s'ajoute, madame la ministre, votre réforme inique

L'AGS est financée par des cotisations patronales et une créance qu'elle prend sur l'entreprise en liquidation ; elle est ensuite remboursée en priorité, ce qui représente environ 25 % de ses ressources. Elle ne coûte donc rien à l'État- il est important de le rappeler. Il est vrai que l'AGS n'est pas parfaite et que sa gestion mérite d'être discutée et débattue. Ce n'est pas un organisme paritaire, puisqu'elle est entièrement administrée par les organisations patronales. Débattons-en ! L'Unédic elle-même, qui en est responsable financièrement, n'a pas de droit de regard sur elle. Discutons-en ! Il est nécessaire de remédier à ces failles, qui sont certaines. Mais au lieu d'ouvrir un débat sur sa transparence ou sa gestion, vous voulez en changer le but initial et ce n'est pas tout à fait la même chose Ce projet de réforme est issu de l'habilitation à légiférer par ordonnance contenue dans la loi Pacte, discutée au Parlement en 2019. Les organisations patronales et de salariés y sont unanimement et fermement opposées, ce qui vaut, en soi, qu'on s'y arrête. Ce projet, nous dit-on, ne serait que la transposition de la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité du 20 juin 2019. C'est là confondre, selon nous, transposition et surenchère, car rien dans cette directive ne concerne l'ordre de priorité des créanciers. Or c'est précisément cet ordre que votre gouvernement se propose de modifier. L'AGS est aujourd'hui prioritaire, et c'est ce qui lui permet de reconstituer sa trésorerie. Cette réforme la verrait passer du troisième au sixième rang des créanciers. Le privilège actuel des salariés se verrait ainsi rétrogradé au profit des frais de justice, donc des administrateurs judiciaires et des banques. Même si, dans une deuxième mouture, vous proposez de ne pas toucher au rang de l'AGS, vous remontez quand même les frais de justice au deuxième rang, donc avant celui de l'AGS, ce qui revient exactement au même S'il existe une difficulté pour payer les frais de justice des administrateurs et des mandataires- là aussi, vous en conviendrez, il faudrait davantage de transparence -, créons un fonds de garantie pour les payer, plutôt plutôt que de déstabiliser tout le système. Les salariés se trouvent une nouvelle fois précarisés et encore davantage soumis aux aléas du marché et à la gestion de leur entreprise, dont ils ne sont aucunement responsables. Ils doivent en être préservés. le Gouvernement opérerait une transformation sérieuse, aux conséquences potentiellement majeures, puisqu'elle porterait atteinte aux fonds propres de l'association, alors que la hausse des dépôts de bilan attendue pour l'automne, avec la fin annoncée des aides publiques, nous enjoint de défendre clairement le superprivilège de l'AGS. Cela pourrait également conduire à une augmentation des cotisations pour les entreprises dans un contexte déjà difficile- elles veux rappeler que l'AGS est déjà affaiblie par l'ordonnance du 20 mai 2020, qui permet de racheter sa propre entreprise en liquidation, l'AGS et Pôle emploi se voyant ainsi contraints de liquider le passif de l'entreprise, y compris pour des groupes comme Mulliez.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet qui nous occupe est particulièrement primordial dans le contexte anxiogène que nous connaissons et je tiens tout d'abord à remercier les auteurs de la présente proposition de résolution pour leur vigilance. En effet, les salaires des entreprises au bord de la faillite doivent continuer à être versés. Or, nous le savons, avec le déphasage des mesures de soutien à l'économie, tandis que s'esquissera la fin de la crise sanitaire, cette question se posera malheureusement avec davantage d'acuité dans les prochains mois. À ce titre, le Parlement ne peut s'en désintéresser. Dans un rare élan d'unanimité, syndicats comme représentants du patronat ont dénoncé l'avant-projet d'ordonnance destiné à transposer la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité et à adapter en conséquence le droit des sûretés. Selon eux, ce projet viendrait déstabiliser notre régime de garantie des salaires, lequel permet d'allouer des avances à plus de 100 000 personnes qui travaillent dans des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure collective. Aussi, cette proposition de résolution traduit une réelle inquiétude, réaffirme un véritable attachement à un pilier de notre tradition sociale et renouvelle un objectif commun : maintenir cet amortisseur social.

peut estimer que sa place dans la récupération est rétrogradée du troisième au sixième rang au profit des frais de justice. Cette rétrogradation pourrait se faire au détriment des salariés et au bénéfice des administrateurs et mandataires judiciaires. Une telle mesure est difficilement acceptable du fait de ses conséquences prévisibles. Avec cette réforme, une perte de 320 millions d'euros est attendue pour cette année, tandis que la hausse des faillites d'entreprises sollicitera fortement la trésorerie de l'AGS. Les solutions sont simples, connues, mais redoutées : il faudrait soit accroître le taux de cotisation patronale, soit baisser le taux de prise en charge des salaires. Si le n'est plus possible et si la garantie des salaires doit être repensée à l'aune de faillites accrues, il convient de renforcer et non pas d'affaiblir l'AGS. mon soutien à une orientation de cette proposition de résolution consistant à envisager l'ouverture de la protection aux indépendants, ces derniers manquant cruellement d'un filet de sécurité.

Dans quelle mesure comptez-vous prendre en compte les recommandations du rapport de René Ricol ? Cette proposition de résolution a le mérite de mettre en avant un mécanisme de démocratie sociale, dont notre pays peut être fier. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre pays est frappé depuis maintenant plus d'un an par une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Les mesures de restriction visant à réfréner l'épidémie ont pesé et pèsent encore sur la santé économique de nos entreprises. À l'heure actuelle, notre économie est sous cloche. Malgré des trous dans la raquette, les mesures d'aide remplissent leur mission. Le nombre de liquidations judiciaires a même reculé de 37 % en 2020. Cependant, ne nous méprenons pas, les effets de ces mesures ne sont que temporaires et artificiels. Nous repoussons l'inévitable. Une fois la perfusion arrachée, il est vraisemblable que de nombreuses entreprises fermeront ou licencieront des salariés. (OFCE) explique ainsi que 175 000 emplois pourraient disparaître à cause des faillites à venir. Pire, selon une étude conduite avec des économistes du cabinet Asterès, le nombre de faillites pourrait augmenter en 2021 dans une On parlerait ainsi de 250 000 emplois menacés. Voilà le drame humain que nous devons anticiper, si nous voulons mieux accompagner et protéger ces Français qui perdront leur travail. Au lieu de cela, le ministère de la justice a d'autres projets en tête. Sûrement l'art du ... Dans ce contexte si singulier, le Gouvernement a trouvé judicieux de mettre sur la table un projet d'ordonnance, qui prévoit de modifier l'ordre des créanciers privilégiés en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, entreprise, faisant passer les salariés après les administrateurs et les mandataires judiciaires. Quel sens des priorités ! Aberrant, mais cohérent pour un exécutif qui compte faire appliquer son inacceptable réforme de l'assurance chômage en pleine crise économique. Avec ce projet d'ordonnance, le Gouvernement réussit l'exploit de réunir l'ensemble des syndicats contre lui : salariés et patronat sont résolument contre.

et conduirait des milliers de salariés dans des situations de détresse financière. C'est d'une seule voix qu'ils demandent le retrait de ce projet d'ordonnance, inopportun et inapproprié dans cette période. Notre régime de garantie des salaires est parmi les plus protecteurs en Europe. Depuis 2010, plus de 2,4 millions de salariés en ont bénéficié, selon le dernier rapport annuel d'activité de l'AGS. Nous avons le devoir de conserver ce régime, et même de l'améliorer. Le superprivilège dont bénéficie le paiement des salaires est plus que jamais nécessaire. Le supprimer reviendrait à amputer les ressources de l'AGS

Sa rétrogradation entraînera donc nécessairement un déséquilibre qui ne pourra être résolu que par deux moyens : la dégradation de la prise en charge des salaires par l'AGS et/ou l'augmentation des cotisations versées par les entreprises. En temps de covid, ces deux options ne sont pas envisageables ! D'un côté, nos entreprises sont aujourd'hui fragiles

De l'autre, il serait inadmissible de toucher à la prise en charge des rémunérations des salariés licenciés en ces temps de crise qui rendent la recherche d'emploi particulièrement difficile. Enfin, selon les syndicats, rien dans la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité ne fonde cette modification de la hiérarchie des créanciers. Le rapport commandé par Matignon le 8 mars dernier et remis le 21 avril confirme nos craintes. René Ricol y conclut que le projet d'ordonnance rétrograderait l'AGS derrière les frais de justice en cas de liquidation judiciaire. Il appelle d'ailleurs à clarifier les règles existantes concernant l'ordre de priorité des créanciers. Il appelle aussi à conserver l'état actuel du droit en cas de liquidation judiciaire, à savoir des créances salariales superprivilégiées, puis le paiement des frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture. C'est tout l'objet de la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui. Parce qu'il partage les craintes des salariés et des chefs d'entreprise et qu'il est conscient des réalités de terrain et des difficultés que subissent salariés et entrepreneurs,

Pour conclure, nous souhaitons attirer l'attention du Gouvernement sur la gestion de l'AGS. Cette dernière est qualifiée par les syndicats de salariés de « boîte noire » dont le patronat fait ce qu'il veut. L'opacité qui l'entoure pose question. Les administrateurs de l'AGS doivent mieux rendre compte de son activité devant le conseil d'administration de l'Unédic. En d'autres termes, il faut plus de transparence et une meilleure prise en considération des syndicats de salariés. à l'heure où la colère sociale se lève contre la calamiteuse réforme de l'assurance chômage, envoyer le signal d'une telle rétrogradation serait une faute politique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi la proposition de résolution portée par notre collègue Bruno Retailleau et le groupe Les Républicains relative à l'avenir du régime de garantie des salaires, dit AGS Créée en 1973 sur l'initiative du Président Georges Pompidou, l'AGS est un dispositif unique en Europe : elle intervient lorsqu'une entreprise, placée en procédure collective, n'a plus les ressources suffisantes pour verser aux employés leurs salaires l'AGS se substitue alors à l'entreprise pour avancer et verser les rémunérations des salariés. L'AGS bénéficie aujourd'hui d'un superprivilège, lui permettant de figurer en haut de la liste des créanciers de l'entreprise et d'obtenir ainsi une garantie sur le remboursement de ses créances, ensuite reversées aux salariés. Or ce système vertueux est aujourd'hui menacé par un projet d'ordonnance, en cours d'élaboration au ministère de la justice, visant à transposer la directive européenne Restructuration et insolvabilité de 2019. Ce projet prévoit de rétrograder le superprivilège du troisième au sixième rang dans l'ordre des créanciers, en faisant passer l'AGS après les banques et les mandataires de justice. de justice. C'est inacceptable ! Quand on est élu de la République, on ne s'en prend pas aux plus fragiles ; au contraire, on les protège ! Or, avec cette réforme, le Gouvernement fait exactement l'inverse, en plaçant les banquiers et les mandataires avant les salariés. Le risque à moyen terme est que l'AGS ne soit plus en mesure de récupérer l'intégralité de ses créances et ne soit donc plus en capacité de verser aux salariés l'intégralité des salaires. Pour remédier à cela, elle serait contrainte de réduire le taux de couverture des salariés ou d'augmenter le taux de cotisation. Rappelons que l'AGS est financée, d'une part, par une cotisation patronale, d'autre part, par la créance que l'AGS prend sur l'entreprise à la place des salariés, provenant notamment de la trésorerie ou de la vente des actifs. Finalement, le Gouvernement prétend qu'il diminue les impôts et les taxes des entreprises, mais, au détour d'une réforme, il augmente leurs charges sans être directement concerné, puisqu'il s'agit de cotisations qui n'entrent pas dans les caisses de l'État C'est la raison pour laquelle la proposition de résolution que nous défendons aujourd'hui s'oppose vigoureusement à l'évolution envisagée par le Gouvernement et propose de préserver le régime actuel de l'AGS. Tout d'abord, la période critique que nous traversons, liée à la pandémie de covid-19, va inévitablement conduire à des faillites d'entreprises, d'autant que le Gouvernement a annoncé, ce qui est logique, la fin progressive des aides pour soutenir l'économie et la fin du fameux « quoi qu'il en coûte ». L'ampleur du « mur des faillites » reste encore incertaine, mais elle pourrait être d'autant plus importante que les aides publiques ont aussi favorisé la survie artificielle de certaines structures qui étaient déjà en mauvaise posture avant la pandémie. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, le tribunal de commerce connaît une forte baisse d'activité depuis un an, mais, lorsque l'on interroge les agents et les juges, on ressent leur inquiétude : tous redoutent le moment où les entreprises cesseront d'être sous perfusion. En 2008, avec la crise des, l'avalanche de défaillances avait mis à mal le régime de l'AGS, qui avait dû doubler le taux de cotisation des entreprises pour le porter à 0,4 %. La situation pourrait être bien pire avec la pandémie de covid-19, car, malgré une baisse de 33 % du nombre d'affaires ouvertes en 2020, les comptes se sont dégradés du fait d'une baisse des cotisations de 9 %, liée principalement au chômage partiel. Pour faire face au pic de faillites, que tout le monde anticipe, sans avoir à augmenter le taux de cotisation, l'AGS a d'ailleurs déjà contracté trois emprunts représentant un droit de tirage total de 1,5 milliard d'euros à rembourser en 2023. qu'il est nécessaire de ne pas fragiliser davantage un système qui joue pleinement son rôle d'amortisseur social et de soutien aux salariés en difficulté. Le calendrier choisi par le Gouvernement est incompréhensible : il était peu opportun de s'atteler à ce dossier en pleine crise sanitaire et économique. Vous nous dites que la loi Pacte impose un délai pour l'ordonnance, mais, une fois de plus, vous auriez dû laisser la main au débat parlementaire ! Les différents interlocuteurs semblent avoir été peu écoutés et tout le monde s'accorde à dire que rétrograder le privilège de l'AGS est un mauvais coup porté aux salariés et à la garantie de leurs droits. La situation d'un salarié qui gagne le SMIC n'est pas du tout comparable à celle d'une banque. Ce salarié a fourni un travail, pour lequel il doit être rémunéré à tout prix. C'est pourquoi l'AGS doit rester superprivilégiée. La proposition de résolution réaffirme justement le caractère fondamental et inamovible du superprivilège de l'AGS. Elle prévoit un élargissement de son champ d'intervention à des mesures de reclassement des salariés et invite Notre proposition de résolution veut aussi en appeler au bon sens. Pourquoi, alors que le système est ingénieux, protecteur et utile, a-t-on besoin de le changer ? On n'entend jamais parler de l'AGS ; c'est donc qu'il fonctionne bien ! c'est un dispositif privé qui n'impacte pas les finances publiques. Le président de l'AGS a bien résumé la situation, en regrettant que « l'on déstabilise un régime socialement généreux et financièrement vertueux ». Pour tenter d'apaiser la situation, le Premier ministre a commandé un rapport à René Ricol. Il vient d'être rendu public : il confirme que la réforme envisagée rétrograde l'AGS derrière les frais de justice et les banques, et il recommande de maintenir le superprivilège des salariés et de maintenir leur protection en cas de faillite. Vous avez indiqué, madame la ministre, que le projet d'ordonnance serait promulgué d'ici à l'été, sur la base des recommandations du rapport. Je veux croire que vous suivrez sa proposition concernant le maintien du superprivilège des salariés. En conclusion mes chers collègues, avec cette proposition de résolution, nous souhaitons envoyer un signal fort de soutien aux salariés de notre pays, touchés durement par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, dont nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur. Nous souhaitons également adresser un signal d'alerte au Gouvernement, pour qu'il ne dénature pas le régime actuel et garantisse le droit des salariés

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Union Centriste tient à

sociales de cette crise sont encore ténues, voire paradoxales. Les dispositifs mis en place par l'État ont été massifs : chômage partiel ; prêts garantis par l'État ; annulation de charges fonds de solidarité. Ces aides ont permis à nos entreprises de tenir durant les mois de confinement, qui, pour certains secteurs, malheureusement, dure encore.

publics, Olivier Dussopt, a annoncé dans la presse, mi-avril, la fin progressive du « quoi qu'il en coûte », avec des conséquences inéluctables sur un certain nombre d'entreprises, et donc de salariés. Le taux de liquidation directe des entreprises après jugement est passé de 66 % avant crise à près de 80 aujourd'hui. Parmi les entreprises touchées, on dénombre une majorité de très petites entreprises, souvent avec moins de cinq salariés. Face à cette situation, qui risque d'empirer dans les prochains mois, il nous faut préserver au maximum le tissu d'emplois. Certaines entreprises ne pourront pas s'en remettre, nous le savons. Malgré les aides de l'État, malgré la mobilisation des chefs d'entreprise, des salariés, il y aura malheureusement de la casse sociale. C'est pourquoi tout doit être fait pour faciliter au maximum la reconversion professionnelle des salariés et leur assurer les meilleures garanties possible. La France s'est dotée en 1973 d'un système intelligent, unique en Europe, qui permet aux employés victimes d'une procédure collective dans leur entreprise de continuer de bénéficier du versement de leur salaire, malgré les menaces de liquidation judiciaire. Ce régime de garantie est aujourd'hui menacé par la transposition

Le projet d'ordonnance soumis à consultation par la Chancellerie nous fait craindre le pire, avec le risque de rétrogradation de l'AGS du troisième au sixième rang dans l'ordre des créanciers. La perte du surprivilège aurait des conséquences directes pour les salariés, ceux-ci étant menacés de ne plus bénéficier du versement de leur salaire jusqu'à la fin de la procédure collective. Le président de l'AGS a fait part de ses doutes quant au bien-fondé de cette réforme, dénonçant notamment un coût pour le régime de près de 300 millions d'euros par an, soit les trois cinquièmes des sommes récupérées en 2020.

Le régime évalue ainsi à 2,5 milliards d'euros le montant des aides à débloquer en 2021, soit près du double de l'an passé. Les conséquences pour l'ensemble de nos territoires ne sont pas minces, près de 98 000 salariés pourraient en bénéficier. Mes chers collègues, certains dispositifs fonctionnent bien dans notre pays. Ne les détruisons pas ! Le régime de garantie des salaires, voulu par le président Pompidou, vient en renfort des aides que la puissance publique peut mettre en place grâce aux cotisations des employeurs et aux créances prises sur la trésorerie ou la vente des actifs de l'entreprise. Dans ce contexte, la proposition de résolution que porte aujourd'hui le groupe Les Républicains est un appel. Appel à ce que soit préservé le régime actuel, qui a fait ses preuves et qui ne coûte pas un centime d'argent public. Appel à ce que soit maintenu le surprivilège dont bénéficie aujourd'hui l'AGS dans l'ordre des créanciers, qui lui permet de remplir à bien ses missions. Appel à ce qu'il soit mis fin, dans la période de difficultés économiques et sociales actuelles, à des réformes hâtives et aux conséquences mal évaluées. Je soutiens pleinement cette proposition que je voterai en pensant à l'ensemble des salariés, des employés de notre pays qui paient au prix fort cette crise. Aux risques de licenciements et de faillites, ne rajoutons pas l'impossibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés méritants la juste rémunération

que les travailleurs soient mieux défendus en pareil cas et qu'ils soient une priorité sur l'actif des sociétés. » Ces mots, prononcés par le président Georges Pompidou en septembre 1973, annonçaient la création de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés qui intervient quand une entreprise se trouve en procédure collective et n'a pas les fonds disponibles pour payer les salaires. Elle se substitue alors à l'entreprise défaillante et prend en charge le versement des rémunérations ou des indemnités de licenciement. L'AGS remplit ainsi le rôle d'un véritable amortisseur social, et nul doute que, dans le contexte actuel de crise sanitaire, cette mission est essentielle. C'est ce que rappelle avec justesse la proposition de résolution de Bruno Retailleau. En contrepartie, l'AGS bénéficie d'un superprivilège et figure parmi les premiers créanciers. Ce mécanisme, unique en Europe, est particulièrement efficace, rapide et ne coûte rien à la collectivité. Vous comprendrez, madame la ministre, que, dans ces conditions, l'avant-projet d'ordonnance préparé par le ministère de la justice ait suscité quelques inquiétudes. Les syndicats et le patronat sont d'ailleurs unanimes- fait exceptionnel ! -pour dénoncer cette réforme, qui menace de rétrograder le remboursement des créances salariales de l'AGS. Certes, les services du ministère avaient réfuté les critiques des partenaires sociaux, mais René Ricol, dans le rapport qu'il vient de rendre à la demande du Premier ministre, confirme leurs craintes. Même si la portée du déclassement doit être relativisée, l'avant-projet rétrograde bien l'AGS dans le classement des créanciers privilégiés, en dépouillant l'institution du superprivilège des salariés. Comme l'a rappelé le président du conseil d'administration de l'AGS, l'équilibre du mécanisme repose sur une cotisation patronale de 0,15 % et la capacité de récupération des avances consenties aux salariés, millions à 500 millions d'euros par an. La rétrogradation entraînerait une perte de 200 millions à 300 millions d'euros en année pleine. Les conséquences, dans une période où le nombre de liquidations risque d'exploser, seraient particulièrement néfastes. Certes, les défaillances sont pour l'instant contenues grâce aux aides publiques pour faire face à l'épidémie de covid. On peut toutefois craindre une augmentation du nombre de faillites en sortie de crise une sollicitation encore plus importante de l'AGS, qui a d'ores et déjà contracté trois emprunts pour pouvoir verser les salaires de 2021 et 2022. Divers instituts économiques estiment ainsi à 45 000 le nombre de défaillances d'entreprises en 2021 et à plus de 60 000 leur nombre pour l'année prochaine. Madame la ministre, pourquoi vouloir ainsi déstabiliser un régime socialement généreux ? Pourquoi organiser la rétrogradation de l'AGS dans l'ordre des créanciers au nom d'une directive européenne qui ne traite pas de cette question ? Pourquoi, surtout, choisir de le faire dans le contexte économique actuel ? Ce projet de réforme va déstabiliser le régime de garantie des salaires en réduisant fortement ses possibilités de récupération des sommes avancées. Ce sont finalement les salariés qui en pâtiront, avec une dégradation de la prise en charge des salaires et des indemnités. La proposition de résolution de Bruno Retailleau et de ses collègues rappelle avec justesse qu'il est plus que jamais nécessaire de préserver notre modèle de protection des salariés. J'y insiste, la crise nous impose de demeurer vigilants pour protéger cet outil, outil, qui a versé 1,5 milliard d'euros à plus de 180 000 salariés en 2019. Je me félicite d'ailleurs des conclusions de René Ricol, qui préconise notamment le maintien du remboursement prioritaire de l'AGS. Ce texte met également en lumière la nécessité de prévoir un mécanisme spécifique de garantie des salaires des indépendants, qui ont été durement éprouvés par la crise. Les difficultés ne cessent de s'accumuler pour ces 3,6 millions de professionnels. Je sais que le ministre délégué aux PME doit, dans les prochaines semaines, préparer un plan visant à renforcer leur protection. Espérons qu'il sera à la hauteur des enjeux. Madame la ministre, je ne peux qu'encourager le Gouvernement à préserver le régime actuel de garantie des salaires, voire à l'améliorer, comme l'y encourage cette proposition de résolution en faveur de laquelle, vous l'aurez compris, le groupe du RDSE votera à l'unanimité.

Monsieur le président, monsieur le président Serge Babary, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai écouté attentivement les observations et inquiétudes des différents orateurs. Je souhaite y apporter quelques éléments de réponse. Avant d'aborder l'avenir du régime de garantie des salaires, je voudrais rappeler les principales mesures de protection des entreprises et des salariés face à la crise. Depuis plus d'un an, la priorité du Gouvernement est et restera de prévenir les défaillances d'entreprises et les destructions d'emplois face au choc économique induit par la crise sanitaire. Prêts garantis par l'État, fonds de solidarité, activité partielle : ces dispositifs exceptionnels sont autant de mesures de soutien économique et de protection des emplois. Le « quoi qu'il en coûte », toutes les travées pourront en convenir, est plus qu'une formule : c'est une réalité ! S'agissant de l'activité partielle, elle bénéficiait encore, au mois de mars, à 2,3 millions de salariés, et sans doute à plus de 3 millions au cours du mois d'avril. Voilà un an, c'est-à-dire au plus fort du premier confinement, ce dispositif de prise en charge des salaires par l'État et l'Unédic concernait 9 millions de salariés. Cette protection bénéficie tout particulièrement à certains secteurs plus touchés que d'autres par les restrictions sanitaires : l'hébergement-restauration, le commerce et le service aux entreprises. Je rappelle que nous avons consacré près de 30 milliards d'euros à ce dispositif l'an dernier, et que nous fléchons plus de 10 milliards d'euros supplémentaires cette année. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont ainsi préservés au sein des entreprises. De ce point de vue, le Gouvernement a pleinement tiré les leçons de la crise financière de 2008-2009. Dans la perspective d'une levée progressive des restrictions sanitaires, nous menons, en compagnie de Bruno Le Maire, des concertations avec les secteurs professionnels et les partenaires sociaux sur l'évolution de ces mesures de soutien. À cela s'ajoute l'activité partielle de longue durée, qui concerne les secteurs dont l'activité est durablement ralentie du fait de la crise. À ce jour, 52 accords de branche ont été conclus, concernant près de 5 millions de salariés. Là encore, le taux de prise en charge des salaires par l'État est élevé pour permettre aux entreprises concernées de rebondir en conservant en leur sein les compétences dont elles auront besoin pour la reprise. Sachez que le Gouvernement prend pleinement la mesure de la situation économique, mais, malgré les mesures exceptionnelles de soutien, nous savons qu'il y aura des mauvaises nouvelles. C'est dans ce contexte qu'intervient la proposition de résolution examinée cet après-midi. Beaucoup a déjà été dit par les orateurs des groupes. Comme il a été rappelé, le régime de garantie des salaires permet, depuis près de cinquante ans, d'assurer à tous les salariés le maintien de leur rémunération pendant les procédures collectives, sans délai d'attente ni période de carence. C'est un régime innovant et socialement protecteur, auquel le Gouvernement est fortement attaché. Il s'agit en effet d'un véritable amortisseur des soubresauts de l'activité économique et de leur impact sur les salariés. Il est financé exclusivement par des cotisations patronales et trouve son équilibre dans la possibilité de récupérer ces avances de salaires en priorité sur les actifs de l'entreprise. Ainsi, il dispose d'un superprivilège par rapport aux autres créanciers de l'entreprise. La réforme du droit des sûretés et la transposition par voie d'ordonnance de la directive Restructuration et insolvabilité de 2019 ont suscité de fortes inquiétudes de l'AGS et des partenaires sociaux. En effet, certains ont pu craindre que le superprivilège disparaisse au profit d'autres créanciers, comme les acteurs mobilisés dans le cadre des procédures collectives : mandataires de justice, avocats, experts. Le projet initial soumis à consultation publique prévoyait d'instituer formellement un rang de classement de priorité des créanciers, faisant redouter une rétrogradation du superprivilège de l'AGS. Or, comme vous le savez, le régime est fragilisé financièrement, puisqu'il a dû emprunter 200 millions d'euros en 2020, du fait d'un montant d'avances net des récupérations supérieur aux cotisations en 2019, c'est-à-dire avant la crise. Par ailleurs, l'AGS pourrait être fortement sollicitée du fait des faillites d'entreprises, qui auraient dû être en cessation de paiements en 2020 ou en 2021, mais qui, grâce aux aides, ont été préservées pendant la crise. La question du rôle et de la survie du régime a donc légitimement été soulevée. Certains se sont émus de la priorité qui serait accordée aux frais de justice, c'est-à-dire au paiement, avant l'AGS, des administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que de leurs conseils, avec un risque de diminution des récupérations. Le sujet n'est pas simple, car, si nous savons que le paiement des salaires est une priorité à l'occasion d'une procédure collective, la survie de l'entreprise en est également une. Or cela nécessite de rétribuer ceux qui travaillent pour la remettre à flot. Dans ce contexte, le Gouvernement a tenu à répondre à l'inquiétude liée à l'évolution du régime de garantie des salaires. Début mars, le Premier ministre a confié à M. René Ricol

Tout d'abord, il convient clairement de réaffirmer le superprivilège de l'AGS et de maintenir son rang de créance. Si la directive a, notamment, pour objectif de simplifier et de clarifier les procédures, elle ne nous interdit pas d'exclure de la liste des créanciers certains d'entre eux, qui, de fait, n'entrent pas en concurrence avec le superprivilège. C'est le cas des administrateurs et mandataires, qui gèrent les procédures et font l'interface avec l'AGS. Pour éviter des frais de justice trop importants, notamment en raison du recours à des experts ou à des avocats, nous mettrons en place, avec le garde des sceaux, des mesures visant à rendre plus transparents lesdits frais et et à mieux les contrôler, sous l'autorité des juges. Cet encadrement, qui, de fait, est dans l'intérêt de tous, permettra à l'AGS de bénéficier d'un droit de récupération plus large. C'est pourquoi nous soutenons votre proposition de résolution sur le volet de la préservation du régime. Les partenaires sociaux devront, par ailleurs, réfléchir à l'évolution des taux de cotisation pour favoriser le retour à l'équilibre du régime. S'agissant des deux autres pistes évoquées, à savoir donner un rôle plus important à l'AGS dans le reclassement des salariés touchés par les procédures collectives et ouvrir le régime aux indépendants, ma position est plus réservée. Certains outils existent déjà pour faciliter le reclassement, comme le contrat de sécurisation professionnelle, qui permet aux salariés dont l'entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire de disposer d'un accompagnement renforcé en cas de licenciement pendant douze mois, avec un maintien de 75 % de la rémunération.

Si, dans la pratique, l'intervention de l'AGS porte uniquement sur des mesures annexes aux formations prévues dans les PSE, par exemple les frais de déplacement pour les formations, il est actuellement possible d'aller au-delà sans qu'il soit nécessaire de modifier son champ de compétences. J'attire toutefois votre attention sur le fait que, si de nouvelles mesures d'accompagnement devaient être financées par le régime, cela pourrait avoir des répercussions financières, et donc impliquer une augmentation des cotisations. S'agissant de l'ouverture du régime aux indépendants, cela conduirait à changer radicalement sa nature. L'AGS garantit une créance salariale et agit en substitution des salariés. Elle dispose en ce sens d'un superprivilège sur les actifs de l'entreprise. Si je comprends parfaitement la détresse de certains indépendants, qui, face aux difficultés de leur activité, se retrouvent sans ressources, le choix d'élargir le régime à cette catégorie de travailleurs conduirait à transformer la garantie salariale en une garantie pécuniaire, et donc changerait la nature du régime. Les pertes de revenus auxquelles doivent faire face les travailleurs indépendants en cas de défaillance de leur entreprise relèvent d'autres mécanismes assurantiels. Pour autant, Alain Griset et moi-même sommes particulièrement attentifs à leur situation économique et sociale et ouverts aux propositions du Sénat pour leur permettre d'accéder à une meilleure protection. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cette proposition de résolution. Monsieur le président Babary, je vous le redis, je reste pour venir présenter les dispositifs de protection de l'emploi et des compétences que nous mettons en oeuvre devant la délégation sénatoriale aux entreprises. La discussion

alors que s'ouvre ce débat, je pense à mes compatriotes qui nous écoutent sur cette terre de Nouvelle-Calédonie, perdue dans le Pacifique et si lointaine vue de Paris. Les uns sont à la recherche d'un chemin vers l'indépendance, les autres ont choisi depuis longtemps celui de la France, mais tous poursuivent leur marche dans les ténèbres, en se cognant contre les murs. Et maintenant, que fait-on ? C'est la question que j'entends vous poser, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Malheureusement, je ne suis pas certain que les réponses abondent. Alors que l'accord de Nouméa est désormais un accord ancien, dont l'esprit est moribond et la lettre sans espoir, personne ne sait comment en sortir, personne ne sait ce qui va se passer. Vous comprendrez donc que cette situation génère une profonde et légitime inquiétude au sein d'une population qui ressent l'impasse dans laquelle elle a été menée. Cette angoisse se double d'une incompréhension

des plus hautes autorités de l'État, comme si la revendication d'indépendance avait plus de légitimité que le combat qu'elle mène pour rester française. Pourtant, depuis trente ans, la Nouvelle-Calédonie est engagée dans un processus exemplaire. Après les violents affrontements des années 1980, qui nous ont conduits à une quasi-guerre civile, nous avons choisi le chemin de la paix et de la réconciliation. En 1988, la signature des accords de Matignon, scellés par la poignée de main de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou, a mis un terme à l'escalade de la violence. Dix ans plus tard, ces accords ont trouvé leur prolongement dans l'élaboration d'une solution consensuelle, qui s'est traduite par la signature de l'accord de Nouméa.

et qu'il nécessitait, pour s'épanouir, de la confiance, de la sérénité et une vraie sincérité, en dehors de toute arrière-pensée, notamment, électoraliste. Je fais le constat aujourd'hui, devant vous, que l'accord de Nouméa a été un acte manqué. Il a été dénaturé dès 2007, avec le gel du corps électoral pour les élections provinciales, qui a justifié par la suite toutes les revendications et toutes les surenchères des indépendantistes. a été géré de manière partisane par tous ceux qui y trouvaient leur intérêt. Il a été confisqué quand on a voulu faire prévaloir son texte sur son esprit. Au lieu de le faire vivre, de le laisser s'épanouir et se transformer, on l'a enfermé, monsieur le ministre, dans une formule coupable, « l'accord, tout l'accord, rien que l'accord », qui empêchait toute évolution. Pendant des années, j'ai proposé de rechercher cette sortie harmonieuse de l'accord, cette nouvelle solution consensuelle, ce nouveau compromis qui aurait constitué la suite et cohérente de ce que nous vivons depuis trente ans et serait venu compléter cet accord imparfait. Mais je n'ai été entendu ni de ma famille politique, ni des indépendantistes, ni de l'État, et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une impasse ! Faute d'être parvenus à un nouvel accord, nous en sommes réduits à l'affrontement sans fin de convictions inconciliables. J'avais aussi la conviction que nous devions faire l'économie de ces référendums mortifères, qui ne pouvaient que raviver les tensions, les divisions et les affrontements. À deux reprises déjà,

et que, quel que soit le résultat, nos convictions et celles des indépendantistes ne varieront pas. C'est aussi un exercice dangereux. Nous qui étions des partenaires, nous sommes redevenus des adversaires, comme si nous n'avions pas travaillé et géré la Nouvelle-Calédonie ensemble, comme si nous n'avions pas porté une ambition commune. Ces référendums à répétition sont devenus un engrenage infernal, qui anéantit toute capacité de dialogue. Je retiens néanmoins deux enseignements de ces consultations. Le premier est qu'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance. Le second est qu'une triple fracture- politique, identitaire et géographique Les électeurs du Sud sont massivement favorables au maintien de la Calédonie dans la France. Les électeurs du Nord et des îles sont massivement favorables à l'indépendance. Nous devons, sans concession, regarder cette réalité en face, même si elle bouscule nos certitudes et nos ambitions. Malgré les efforts de rééquilibrage financiers et les initiatives économiques, culturelles et sociales, nous n'avons pas progressé dans la construction d'une communauté de destin. Les indépendantistes sont et resteront farouchement indépendantistes ; quant à nous, nous sommes et nous resterons indéfectiblement attachés au maintien de la Calédonie dans la France, parce que chacun de nous reste et restera intimement attaché à son identité. Ces référendums auront malheureusement enfermé la vie politique locale dans une logique d'affrontements identitaires. À l'évidence, ce que nous avions imaginé il y a vingt est dépassé. La réalité est que la Nouvelle-Calédonie est une terre aux identités multiples, où chacun doit pouvoir développer ses atouts dans une relation saine, stable et pérenne. la recherche à tout prix de convergences factices nous a conduits à des confusions néfastes. La réalité est que nous avons un défi à relever apprendre à savoir vivre ensemble, assumer nos différences pour rendre notre collectivité humaine plus forte, et nous entendre sur nos divergences pour en limiter les effets. Je crois que nous en sommes capables.

Au-delà de la formule, qui peut sembler un bel oxymore, négocier un désaccord, c'est l'assurance d'une coexistence apaisée, dans le respect de nos identités et de nos différences.

afin d'en limiter les effets, de reconnaître ce que nous partageons, d'accepter ce qui nous sépare et, sur cette base, d'organiser notre avenir. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de tracer devant vous les grandes lignes de cette solution ; j'espère qu'elle permettra à la Calédonie d'inventer son avenir

le second, à réaffirmer la prééminence de la collectivité provinciale. Quand je dis qu'il faut avoir cette terre de Calédonie en partage, je pense à cette nuit interminable de juin 1988, alors que nous posions les principes fondateurs des accords de Matignon, lesquels, en partageant le territoire en trois provinces, ont permis le retour à la paix civile. Personne, jusqu'à aujourd'hui,

C'est donc sur cette base retrouvée que je propose d'unifier en harmonisant les contraires, au lieu d'uniformiser en écrasant les différences. Le coeur de cette proposition, c'est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. conséquence, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de trois provinces dotées de la compétence de principe et garantissant les différentes identités de la Nouvelle-Calédonie. Les communes seront des collectivités des provinces et certaines compétences pourront leur être déléguées. Chaque province sera dotée de son conseil coutumier kanak, composé de représentants des chefferies des aires coutumières de son ressort. Surtout, chaque assemblée de province sera sera élue selon son propre régime électoral afin que nul ne soit exclu. L'État continuera à assurer toutes les compétences régaliennes- défense, justice, ordre public, monnaie, affaires étrangères mais les provinces pourront partager certaines de ses prérogatives, en accord avec lui. Pour assurer la gouvernance de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, et pour éviter de tomber dans les travers et les lourdeurs du gouvernement collégial mis en place par l'accord de Nouméa, je propose la constitution d'un collège médiateur, composé du représentant de l'État, évidemment, et de représentants des assemblées de province. Son président représentera la Nouvelle-Calédonie en toutes circonstances. Cette gouvernance est un processus de coordination des provinces et de l'État en vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement, mais c'est aussi un mode d'organisation qui impliquera des négociations permanentes, sur un pied d'égalité, entre les provinces. Il s'agira non plus de dicter des priorités mais de se contenter de réguler et d'arbitrer, afin d'assurer le libre épanouissement des provinces. Il s'agira d'une répartition plus horizontale du pouvoir. Le savoir vivre ensemble nécessitera des règles communes, mais, au lieu d'être imposées d'en haut, les mesures prises résulteront d'un processus d'élaboration collective guidée par la recherche de réponses aux défis communs, conformément à des valeurs contenues dans une charte. définira un engagement de valeurs partagées, de droits et de libertés garantis par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel de la République. Elle exprimera par ailleurs l'adaptation du droit civil aux identités plurielles de la Nouvelle-Calédonie concernant les personnes, la famille, les rapports entre les personnes et leurs rapports au groupe social. Cette solution institutionnelle sera bien sûr soumise à l'approbation des populations intéressées. j'entamais mon propos en évoquant le sort de mes compatriotes qui continuent de cheminer dans les ténèbres. Il est vrai que cela est dû, en grande partie, à cet État que vous incarnez aujourd'hui,

Se débarrasser de la question calédonienne, c'est laisser entendre qu'une indépendance en association ou en partenariat reste possible, à la condition, bien sûr, que les intérêts économiques et militaires de l'État soient garantis. Se débarrasser de la question calédonienne, c'est malheureusement abandonner toute cette population à son sort et alimenter les tensions.

C'est réussir à conjuguer respect de la démocratie locale, respect des identités, respect des différences et intérêt de la France. Monsieur le président, mes chers collègues, je m'adresse à vous car la Nouvelle-Calédonie ne peut plus attendre. Elle a besoin de développer un autre visage. Elle a besoin que, sans attendre, une main lui soit tendue. En incarnant la bonne volonté de la République à l'endroit de tous les Calédoniens, en employant sa culture de la sagesse à résoudre une question territoriale qui peut avoir des conséquences importantes, y compris dans d'autres territoires ultramarins, notre Haute Assemblée pourrait incarner cet espoir et permettre à la Nouvelle-Calédonie de devenir un laboratoire de l'adaptation républicaine aux réalités des territoires et de vivre les différences sereinement. En favorisant par l'intelligence collective la coconstruction d'une solution d'aujourd'hui, nous passerions d'une logique de centralisation, puis de décentralisation, à une logique de regroupement des territoires. Monsieur le président, je veux conclure en vous priant d'avoir en tête le sort du jeune indépendantiste par solidarité identitaire et celui de son ami loyaliste à l'identité culturelle si différente. Je vous demande, pour eux, de vous engager afin de les libérer de la peur de l'autre, afin de leur permettre d'être français ensemble, en valorisant respectant leurs différences et en inscrivant leur avenir dans une appartenance commune. La parole

Alors que nous arrivons au terme du processus de Nouméa, le Caillou a occupé, occupe et occupera votre gouvernement, monsieur le ministre, comme aucun autre au XXI siècle. Il sera également l'un des premiers gros dossiers du gouvernement qui sortira des urnes en 2022. La demande d'un troisième référendum d'autodétermination intervient dans une situation économique dégradée, dans une situation politique fragmentée et dans une situation sociale toujours plus conflictuelle. Cela n'a rien d'étonnant, alors que l'on s'approche de la fin d'un processus qui a été entamé il y a plus de trente ans et dont l'issue représente un vide politique, une feuille presque blanche qui reste à écrire. La situation particulièrement tendue et bloquée de l'hiver dernier a néanmoins connu une légère accalmie. Je salue à ce propos l'intervention bienvenue de l'État, qui a favorisé une solution de reprise du complexe minier Vale.

Rappelons que ce site accueille la plus grosse usine mondiale d'acide sulfurique, dans une zone riche d'une biodiversité exceptionnelle. Vous vous doutez bien que les écologistes seront particulièrement exigeants sur ce dernier point. Ce week-end, c'est la paralysie politique qui durait depuis la mi-février qui semble trouver une issue, avec le compromis qui s'esquisse entre les formations indépendantistes à la tête du gouvernement de l'île. Entre-temps, la demande d'un troisième référendum, à l'automne 2022, a été effectuée. Vous avez invité toutes les formations politiques calédoniennes à Paris à la fin du mois, monsieur le ministre, pour envisager ce référendum et les conséquences des deux scénarii dans lesquels la Nouvelle-Calédonie pourrait s'engager à l'issue de ce scrutin. Votre démarche nous semble la bonne. Néanmoins, elle ne sera utile que si toutes les forces politiques sont effectivement présentes. Aussi, il nous paraît essentiel de convaincre les partis indépendantistes de faire le déplacement, en affinant rapidement votre programme de travail et, au besoin, en envoyant un émissaire gouvernemental sur l'île pour caler les choses. Sans cela, vous ne parviendrez pas à tenir votre promesse d'un travail consistant sur les conséquences du oui et celles du non, un travail à même d'éclairer le débat référendaire, les électrices et les électeurs, mais aussi tout le pays. Le calendrier étant ce qu'il est, vous ne pourrez pas vous engager sur une gestion de l'après-référendum, qui ne sera peut-être pas du ressort de l'exécutif actuel. Nous vous demandons donc de construire en amont, avec toutes les forces politiques nationales, le compromis politique le plus large possible sur ce que sera l'attitude de la France. pourra soutenir et favoriser, en cas de victoire du non, l'émancipation du peuple kanak, seule à même d'apaiser les tensions, ou bien accompagner l'indépendance, en cas de victoire du oui, autant qu'il le faudra et dans les meilleures conditions possible. C'est la seule manière d'apporter des perspectives relativement stables aux Calédoniens, pour un débat transparent qui ne courre par le risque d'une spectaculaire volte-face à la fin du printemps 2022. Quel que soit le choix du peuple calédonien, il n'effacera pas l'héritage colonial de l'île ni son corollaire de divisions, d'inégalités socioéconomiques inacceptables et de conflictualité. Quel que soit ce choix, il ne réglera pas la trop forte dépendance de l'île envers l'extraction du nickel, aux très graves conséquences écologiques et sociales. Quel que soit ce choix, il ne fera pas disparaître l'intérêt, parfois presque prédateur, de la France pour l'île, qu'il s'agisse de ses ressources minières où de l'intérêt géostratégique de sa présence dans le Pacifique. La dépendance envers la métropole qui s'est construite depuis plus d'un siècle est de toute façon beaucoup trop forte pour permettre au peuple calédonien de disposer librement de lui-même. Les destins de la France et de la Nouvelle-Calédonie resteront liés, quel que soit le choix des urnes. Mais pour favoriser autant que possible un choix autonome, la France doit apporter des garanties sur le devenir politique de l'île, quel que soit le scénario choisi démocratiquement dans dix-huit mois. Monsieur le ministre, c'est une tâche exaltante à laquelle vous vous attelez : contribuer à inventer le devenir d'un territoire et de ses populations pour se libérer enfin du poids de l'héritage colonial et pour engager une transition sociale, économique et écologique à même de réduire les inégalités,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est humblement, en tant que sénateur des îles Wallis et Futuna, connaissant à ce titre le tiraillement entre deux cultures, que je me tiens devant vous aujourd'hui. C'est également en tant qu'Océanien français, profondément ancré dans les traditions et les coutumes de mes îles, que je prends la parole pour témoigner comme voisin et spectateur privilégié de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, surnommée « le Caillou ». À cette occasion, je salue chaleureusement la communauté wallisienne et futunienne de Nouvelle-Calédonie. Celle-ci entre dans la dernière phase d'un processus inédit, inédit, qui a été une source exceptionnelle d'optimisme. Il a démontré la capacité des femmes et des hommes à trouver, au sein de la République française, des solutions novatrices pour répondre aux défis qui s'imposent à eux. Toutefois, cette source se tarit à mesure que se rapproche le prochain référendum. Mes chers collègues, ne nous voilons pas la face sur la situation de la Nouvelle-Calédonie ! Ce territoire reste divisé entre deux communautés. Si elles s'acceptent et se respectent désormais, elles continuent toutefois de nourrir des ambitions antagonistes pour leur avenir. Les inégalités y sont encore trop fortes, d'autant qu'elles s'inscrivent dans une réalité ethnique qui les rend révoltantes et insoutenables. D'un côté, les indépendantistes militent pour que la communauté kanake, dont chacun sait ici les souffrances et les humiliations qu'elle a subies dans son histoire, recouvre une dignité et une légitimité existentielles qui lui sont dues, avec comme horizon l'accession de la Nouvelle-Calédonie à son indépendance. De l'autre, les loyalistes, attachés aux valeurs françaises et à l'accompagnement de l'État, aspirent à évoluer en restant au sein de la République. Cette division est partagée de manière proportionnelle par l'ensemble des différentes communautés vivant sur le Caillou ; les deux premiers référendums en sont le reflet. Par deux fois déjà, les Calédoniens et les Calédoniennes ont prouvé leur capacité à se réinventer en faisant le pari de l'intelligence collective, au détriment de l'affrontement. Cela a été symbolisé par la poignée de main historique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Les Calédoniens seront donc bientôt amenés, une fois encore, à décider de leur avenir institutionnel. Au nom des Français que nous représentons, je veux leur dire combien nous souhaitons qu'ils fassent le choix du dialogue et de la sagesse. Mes chers collègues, la Nouvelle-Calédonie est à l'orée d'une nouvelle période de son histoire. Elle fait cependant face à d'importants défis. En tant qu'île du Pacifique, elle sera aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique, comme l'ensemble des terres d'outre-mer menacées par la montée des eaux. Elle doit également composer avec des perspectives économiques moroses. L'économie calédonienne reste dépendante d'un or vert et d'usines non rentables, qui n'ont pas tenu leurs promesses de diversification, malgré l'intervention de l'État. Nichée au coeur de l'axe indopacifique, sur lequel le président Emmanuel Macron a eu raison de porter un regard attentif, la Nouvelle-Calédonie attise les convoitises. Ses ressources minières et halieutiques aiguisent l'appétit d'influences dont l'intérêt pour les droits humains et écologiques est bien moins marqué que celui de la France. Comment la Nouvelle-Calédonie compte-t-elle répondre à tous ces défis ? Comment compte-t-elle financer la diversification de son économie ? Comment compte-t-elle assurer le rééquilibrage économique et social ? Comment compte-t-elle résister à la présence croissante d'influences étrangères ? Enfin, quelle sera la stratégie géopolitique de la France dans la région ? autant de problématiques qui seront au centre des discussions dans les semaines à venir, grâce à l'implication du ministre Sébastien Lecornu, que je salue. Il est urgent d'échanger sur les conséquences du oui et du non. C'est un impératif absolu. Mais la principale question, mes chers collègues, est la suivante quelle est la position de l'État français dans ce débat ? Si l'avenir de la Nouvelle-Calédonie n'a pas vocation à se dessiner dans les hémicycles métropolitains, il est néanmoins indispensable que l'État et la représentation nationale prennent toute leur place dans ce débat. En engageant l'avenir des Calédoniens, le Gouvernement engage également celui des Français. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier le président Larcher d'avoir pris l'initiative de cet échange porteur d'espoir.

À quelques mois du prochain référendum, aucun accord n'a été trouvé. Aucune assurance n'est donnée aux Calédoniens, qu'ils soient pour ou contre l'indépendance. Pour ma part, j'invite les leaders et dirigeants calédoniens à une concertation collective, je les invite à penser de nouvelles perspectives et des garanties susceptibles de rassurer la population dans son ensemble. Le débat calédonien interroge tous les Ultramarins, mais également chaque Français. Il soumet à notre réflexion l'évolution des rapports que nous, collectivités ultramarines, pouvons entretenir avec la métropole. Cette relation se doit d'être apaisée, la place et les coutumes de chacun doivent respectées. Elle doit aussi être pérenne, pour lever le voile de l'incertitude et permettre à tous de se projeter vers un destin commun. Enfin, elle doit offrir à notre jeunesse les moyens de réussir à relever les nombreux défis qu'elle devra affronter. Cette jeunesse nous écoute, à Nouméa, à Koné, à Wé, mais aussi à Mata-Utu, à Saint-Denis, à Pointe-à-Pitre ou à Papeete. Elle porte nos espoirs, même dans des situations compliquées, comme quand elle doit venir étudier en métropole. Mais cette jeunesse n'abandonne pas : elle nous regarde avec insistance. Aujourd'hui, elle attend, comme tous les Calédoniens, que ses représentants et l'État soient clairs sur l'avenir que nous lui préparons. Pour cela, nous devons dire les choses. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement doit rassurer les Calédoniens et les Français. Les silences de cet horizon incertain poussent chacun dans ses derniers retranchements et creusent le lit d'une inquiétude et d'une colère dont on sait qu'elles seront à l'origine de tragiques événements. Il est de notre responsabilité de faire maintenir le dialogue entre les différentes composantes calédoniennes, afin que la dernière consultation aboutisse à un avenir radieux et prometteur pour l'ensemble des Calédoniens.

de la France d'outre-mer, soulignait que, un siècle plus tôt, la France adoptait la Nouvelle-Calédonie en affirmant des droits sur cette terre, il savait aussi que ces droits comportaient des devoirs. C'est à l'un de ces devoirs que nous sommes d'autant plus confrontés que, pour notre part, nous estimons que la Nouvelle-Calédonie a pleinement sa place dans la République.

à son terme. Le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie est le fruit d'une histoire coloniale souvent pesante et d'un processus de décolonisation laborieux. Depuis les accords de Nouméa jusqu'au troisième référendum, qui pourrait avoir lieu d'ici à 2022, nous demeurons à la recherche d'un équilibre avec ce territoire aux antipodes de la métropole. Les enjeux politiques et sociaux y sont particulièrement complexes et justifient pleinement qu'un débat soit consacré à ces questions, pour lesquelles chacun doit savoir faire preuve de prudence et de tempérance. D'autant que la recherche d'équilibre se traduit également par des aspects précis et délicats, notamment d'un point de vue juridique. Je souhaite évoquer en particulier l'équilibre de l'application, en Nouvelle-Calédonie, de deux régimes de droit inhérents, si l'on schématise, à l'existence de deux populations : celle des autochtones kanaks et celle qui résulte du processus colonial. Comme nous le savons, une partie du droit kanak originel continue d'être appliqué, notamment par le truchement du statut civil coutumier. De ce point de vue, la coexistence des systèmes juridiques et normatifs pose des difficultés concrètes. la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui a suivi les accords de Nouméa, est venue organiser l'articulation des droits coutumiers et du droit commun. Il n'en reste pas moins que les dispositions de cette loi ne résolvent pas pleinement les questions pratiques qui se posent aux autorités coutumières. Leur complexité est telle que les quelques articles de notre législation permettent mal aux juridictions de faire face à ce que l'on peut qualifier d'une crise de juridicité de la coutume. Voilà donc l'une des problématiques fondamentales à laquelle se confronte la sortie des accords de Nouméa. En plus des enjeux politiques et institutionnels, le choix de l'indépendance ou du maintien devra aussi tenir compte de cette dimension juridiquement concrète. Quelle que soit la solution retenue, qu'adviendra-t-il du droit commun, du droit coutumier et de ce qui a déjà été acquis dans leur articulation ? Certaines avancées ont déjà eu lieu. Ainsi, le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a adopté, en 2011, une délibération sur un cadre de résolution des conflits en milieu coutumier, qui vise à s'appliquer avant que le conflit ne dépasse le terrain coutumier pour gagner le terrain judiciaire et pénal. Il reste néanmoins du chemin à parcourir pour aboutir à un système pérenne, que soit choisie la voie du maintien ou celle de l'indépendance. Par ailleurs, si essentielle soit-elle, cette question de l'indépendance tend parfois à mettre un voile sur d'autres difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie. Je pense, par exemple, à certaines problématiques matérielles liées aux infrastructures du réseau routier, qui ont souffert et souffrent toujours du passage de la dépression tropicale Lucas au mois de février dernier. Durant plusieurs mois, des routes furent barrées ou endommagées, compliquant significativement la vie quotidienne de nos concitoyens. Les services techniques sont débordés et peinent encore à répondre à toutes les demandes. Je n'évoque pas ces questions par goût de l'anecdote, mais parce qu'elles sont susceptibles d'affecter la qualité du débat démocratique engagé depuis plusieurs années et qui devrait se poursuivre encore. Je veux souligner d'ailleurs que le Sénat doit prendre toute sa place dans le processus. Nous devrons rester mobilisés pour nous prononcer sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie après les échéances que nous connaissons. Au fond, le choix de l'indépendance ou du maintien dans la France ne suffira pas à résoudre certaines difficultés structurelles et économiques. Les référendums ne réparent pas les routes et les ponts ; se rendre aux urnes ne suffit pas à éteindre les difficultés ... Aussi, je conclurai mon intervention en formulant le souhait que la France, tout en respectant l'expression démocratique dans laquelle le Gouvernement est pleinement investi- je m'en félicite -, poursuive son soutien à la Nouvelle-Calédonie afin que cette dernière accède à davantage de sérénité tant politique, qu'économique et sociale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est marquée par des épisodes douloureux, par des tensions qui ont abouti aux « événements » des années 1980, quasi-guerre civile qui a fait couler le sang entre partisans et opposants à l'indépendance. C'est dans ce contexte de violence qu'ont été signés les accords de Matignon en 1988, puis l'accord de Nouméa en 1998. À strictement parler, nous arrivons au terme du processus référendaire, puisque les indépendantistes du Congrès ont demandé la tenue du troisième référendum. D'ici à octobre 2022, la préparation du dernier référendum ne peut se limiter à la seule réponse binaire d'un oui ou d'un non à l'indépendance.

Le précédent référendum a été la scène d'une campagne très violente entre indépendantistes et loyalistes. Ces derniers ont récemment perdu le contrôle du Gouvernement, alors qu'ils y étaient majoritaires depuis 1998. Le dialogue engagé par l'État entre l'ensemble des interlocuteurs est essentiel, car, quoi qu'il arrive, ils doivent faire société. Les conflits politiques créent des situations de blocage institutionnel, comme nous le voyons avec la difficulté pour le nouveau Gouvernement calédonien d'élire son président. L'avant-référendum implique donc une large campagne d'informations et de concertations. D'une part, il s'agit d'expliciter à chaque citoyenne et citoyen calédonien les enjeux liés à ce référendum en matière fiscale, agricole et industrielle, sur la citoyenneté et sur les questions régaliennes nécessaire de recueillir leur avis. Tout en conservant sa neutralité, l'État a ici un rôle à jouer pour mettre ces informations à disposition. Monsieur le ministre, où en est-on dans les consultations lancées à l'échelon Selon l'économiste Olivier Sudrie, si la Nouvelle-Calédonie était un pays indépendant, elle serait la deuxième nation la plus inégalitaire de L'héritage colonial structure encore la société calédonienne avec des disparités ethniques importantes, malgré la division par deux des inégalités entre Kanaks et Caldoches en vingt ans. Le taux de pauvreté de la province Nord demeure de 35 %, contre 9 % au Sud. Il s'élève à 52 % dans les îles Loyauté, où les Kanaks sont encore plus présents que dans le Nord. Les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie huit fois plus élevé que les 10 % les plus modestes. Ces clivages nourrissent la volonté d'indépendance, mais on ne peut affirmer que celle-ci permettrait une réduction des inégalités. Si le oui l'emporte, il nous faudra accompagner les Calédoniens dans leur transition vers l'indépendance et développer la coopération, afin de nous assurer que la dépendance actuelle vis-à-vis de la métropole ne creuse davantage les inégalités. Si le non l'emporte, de nouveaux outils devront permettre de favoriser un développement égalitaire de l'archipel. L'État n'a pas su préserver les identités des différentes populations qui le composent ni faire cesser les discriminations raciales ou reconnaître à leur juste hauteur la place des populations kanakes. Ces lacunes ont créé des incompréhensions ; elles nourrissent les distensions- le prochain référendum n'y mettra pas fin. La démocratie parlera ; nous écouterons le choix des Calédoniens. Mais comment imaginer une destinée commune avec de telles inégalités économiques et sociales ? Le statut juridique n'est pas l'alpha et l'oméga, contrairement à l'objectif de faire fonctionner une société pluriethnique et pluriculturelle. L'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie sont liés par une douloureuse histoire. Que l'archipel demeure dans notre République ou à ses côtés, l'État ne peut s'en déresponsabiliser. À cela s'ajoutent des enjeux d'autonomie économique, l'archipel bénéficiant de ressources qui ne sont aujourd'hui pas mises à profit, comme sa faune et sa flore marines. La dépendance à l'industrie du nickel, qui emploie un salarié du privé sur quatre, dont 60 % d'ouvriers, a montré ses limites, comme l'a prouvé la vente de l'entreprise Vale. Des impératifs non seulement économiques mais aussi environnementaux impliquent une diversification de l'économie calédonienne.

mais ouvrir mon intervention par ces mots de Louise Michel, envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie en 1873 pour avoir été communarde : « Chacun cherche sa route ; nous cherchons la nôtre et nous pensons que, le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux ».

ils étaient 111 : 111 Kanaks exhibés lors de l'exposition universelle de 1931 au parc de Vincennes. On les avait exposés, à côté des crocodiles, parce que les « sauvages » devaient être aux côtés des bêtes sauvages. La brochure disait : « Venez voir les Kanaks, car c'est une race qui va bientôt disparaître. Seul. Il a pris une balle seul, sur la propriété de ses parents. C'était une belle journée de janvier 1985. Il avait 17 ans et la mort a frappé,

C'était deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 1988. Ils étaient 2. Ils venaient pour la levée de deuil, un an après : 2 à serrer les mains, à saluer les autorités coutumières et les familles, quand ils ont été abattus par l'un des leurs. Ils s'appelaient Jean-Marie et Yéyé. C'était un 4 mai. Si je raconte cette histoire, c'est parce que c'est la mienne. Celle d'un Kanak originaire de la tribu de Poindah, dans l'aire coutumière Paici-Camûki, en province Nord. Si je raconte cette histoire, c'est parce que c'est celle de mon peuple, le peuple calédonien. Si je raconte cette histoire, c'est parce que c'est la nôtre, celle de la France. C'est 170 ans d'une histoire dont nous sommes les héritiers. Je prononce ces mots avec gravité, à la veille d'un double anniversaire hautement symbolique, celui de l'assaut de la grotte de Gossanah à Ouvéa et de la signature de l'accord de Nouméa. Mes chers collègues, nous n'écrirons pas sur une page blanche au moment où le peuple calédonien sera appelé à décider, pour la troisième fois en quatre ans, si la Nouvelle-Calédonie doit devenir indépendante ou si elle doit demeurer au sein de la République française. Pourtant, je crois plus que jamais au destin commun entre la France et la Nouvelle-Calédonie, un destin commun nourri par une histoire, une langue, une école et des valeurs, mais aussi par trente ans de souveraineté partagée. Je crois plus que jamais au destin commun du peuple calédonien, lié par des sangs mêlés, une culture métissée et des mémoires entrelacées, ainsi que par une gouvernance partagée des institutions du pays, entre indépendantistes et non-indépendantistes. C'est parce que ces destins communs sont au coeur de notre histoire que je ne veux pas d'un troisième référendum binaire : comment la moitié de la population du pays pourrait-elle imposer son choix à l'autre moitié, quand on connaît notre histoire ? C'est pourquoi nous proposons de substituer à cette troisième consultation un référendum de rassemblement. Construire un référendum de rassemblement, c'est admettre, pour les indépendantistes, que l'indépendance n'est pas une baguette magique face aux inégalités, à l'échec scolaire et à la délinquance qui mine notre société. Construire un référendum de rassemblement, c'est accepter, pour les non-indépendantistes, de revisiter notre lien à la France. Un référendum de rassemblement, c'est conjuguer ce qui nous a jusqu'alors opposés : la souveraineté et la République. Ce sont ces deux essences que nous devrons fusionner pour poser le nouveau poteau central de la grande case du pays. La souveraineté, parce qu'elle est nécessaire en termes de reconnaissance et de dignité pour les indépendantistes, après 170 ans d'histoire. La République, parce qu'elle assure le lien entre toutes les communautés du pays, parce qu'elle nous protège en garantissant notre sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, parce qu'elle nous permet de bénéficier de l'un des niveaux de vie les plus élevés de la région Pacifique. Construire un référendum de rassemblement, c'est conjuguer le oui et le non pour tisser un nouveau consensus sur un avenir partagé, comme lors des accords de Matignon et de Nouméa. Construire un référendum de rassemblement, c'est poursuivre la trajectoire de notre émancipation, tout en restant protégé par la France. Le dialogue prochain, sous l'autorité du Président de la République, pourrait nous offrir cette opportunité. Soit nous sommes capables de poser les bases de ce référendum de rassemblement et son organisation en septembre 2022 fait sens, car elle nous donne le temps de finaliser un projet d'avenir partagé, soit nos échanges sont infructueux et, dans ce cas, autant organiser le troisième référendum dès la fin de l'année 2021, afin d'ouvrir le plus rapidement possible les discussions sur l'après-accord de Nouméa. Mais attention : les discussions après le troisième référendum seront compliquées, car il y a aura alors un vainqueur électoral et un vaincu. Les concessions réciproques pour construire un consensus sont possibles avant le troisième référendum. Après, elles seront très difficiles, voire impossibles. En cas de non, le droit à l'autodétermination devra, de toute façon, continuer à s'exercer. Jusqu'à quand ? Avec quelles conséquences ? Sur ce chemin, certains brandissent désormais comme solution la « partition » du pays ou ses déclinaisons- l 'hyper-provincialisation et la différenciation. Cet apartheid géographique nous conduirait à effacer 150 ans d'histoire commune : les Kanaks avec les Kanaks, les autres avec les autres. Croyez-moi, beaucoup de ceux qui aujourd'hui vivent en province Nord, d'où je suis originaire, sont radicalement opposés à cette perspective Notre réalité, c'est un pays un et indivisible, dont l'accord de Nouméa a exclu, dès l'origine, toute partition en fonction des résultats du référendum. Notre réalité, c'est un pays qui n'a pas de frontières. Le découper, c'est l'amputer, c'est le ghettoïser. Notre avenir, c'est de continuer à conjuguer nos deux rêves pour une même terre, et non et non d'affecter chaque rêve à une terre. C'est, selon moi, le seul chemin possible pour favoriser l'émergence d'un pays rassemblé, en paix avec lui-même et confiant en sa destinée. vive un référendum de rassemblement avec tous les Calédoniens, vive le peuple calédonien, vive la France

Monsieur le président, Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà eu l'occasion de débattre du devenir de la Nouvelle-Calédonie dans des circonstances autrement plus dramatiques. Nous pouvons nous féliciter de ce que ce débat se déroule aujourd'hui dans un contexte de paix civile. Il constitue l'occasion- j'en remercie le groupe LR -d'évoquer le passé, mais surtout l'avenir, à l'aube du troisième référendum sur l'indépendance. Le passé, c'est la colonisation, qui a entraîné un traumatisme durable pour la population d'origine. C'est une histoire qui a vu les Kanaks devenir minoritaires dans leur propre pays. La Nouvelle-Calédonie charrie encore la mémoire de révoltes écrasées dans le sang et de luttes, parfois instrumentalisées, entre les tribus. Malgré ces souffrances indicibles, les Kanaks ont accepté de reconnaître que les femmes et les hommes qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie, qui ont contribué à son développement et à l'effort collectif, ont sans nul doute vocation à participer à la détermination d'un destin commun. C'est ce constat qui figure dans le préambule de l'accord de Nouméa de 1998, accord dans lequel nous nous inscrivons : « Ni nous sans vous, ni vous sans nous » ... Dans le prolongement et la fidélité aux accords de Matignon de 1988, nous sommes tous là dans le même bateau. Ces accords ont durablement instauré un esprit de dialogue entre les signataires. On a beaucoup parlé à l'époque de « miracle » à leur propos, mais ils sont surtout le résultat de la générosité, de l'intelligence, de la détermination d'hommes et de femmes dans un contexte où la violence avait atteint son paroxysme lors de la prise d'otages d'Ouvéa et de son issue sanglante. Ce fut l'honneur des gouvernements Rocard et Jospin, mais aussi de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ainsi que de celles et ceux qui s'inscrivirent dans leur sillage, d'avoir su entendre les revendications du peuple kanak et les doutes des autres composantes de la société calédonienne. Ils ont prouvé que l'État n'est pas seulement autoritaire et répressif, mais qu'il joue d'abord un rôle de pacification. Tout ce qui a été entrepris depuis en Nouvelle-Calédonie repose sur un idéal de tolérance et de respect de l'autre, qui permet d'envisager le passage d'un destin communautaire et parcellaire à la construction d'un destin commun et partagé. Il s'agit maintenant de rester fidèle à ces principes, de garantir le maintien des conditions de la concorde et de la paix.

Il nous revient d'appréhender les conséquences concrètes de tous les scénarios. L'État, sans se départir de son impartialité, laquelle est d'ailleurs garantie par les accords de Matignon, doit s'engager sur la Nouvelle-Calédonie d'après. Ce qui doit primer, c'est d'avoir un processus, un cheminement, qui puisse rassembler. L'État devra proposer une solution, il devra dire comment il accompagnera la Nouvelle-Calédonie dans les voies qu'elle pourra choisir. Aujourd'hui, monsieur le ministre, la voix du Gouvernement doit être plus ferme. Dans ce cadre, nous ne partageons pas ce que suggère notre collègue Pierre Frogier, lui qui fut pourtant l'homme des deux drapeaux côte à côte. Comment peut-il raisonnablement penser que la solution soit le « chacun chez soi », un drapeau au Nord, un autre au Sud. La différenciation politique qu'il propose rime avec confédération.

n'est rien d'autre qu'une partition territoriale à laquelle nous ne pouvons pas adhérer. Cette idée de provincialisation consiste en réalité à accroître les prérogatives des provinces. Ce qui est présenté comme une décentralisation est en fait une division stricte du territoire avec des fortunes économiques particulièrement déséquilibrées.

Il se pose en garant de l'esprit de Nouméa, en refusant fermement la partition et en rappelant que l'héritage Rocard-Jospin est celui d'hommes et de femmes qui ont compris que tout était à redouter si chacun persistait à s'isoler. Faisons place, mes chers collègues, à une nouvelle imagination. Pourquoi ne pas imaginer une solution de dialogue et de compromis, qui pourrait être acceptable en préconisant la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un partenariat institutionnel avec la France ? Elle impliquerait l'inscription d'un partenariat dans les constitutions respectives de chaque pays. Il s'agit en quelque sorte d'une formule d'États associés, qui a déjà fait ses preuves ailleurs dans le monde.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les enjeux liés à la Nouvelle-Calédonie me sont chers et familiers, parce que je m'y suis rendu récemment, comme un certain nombre d'entre vous, parce que mon frère y est installé depuis trente ans- il a travaillé dans les trois provinces et se trouve aujourd'hui responsable de la vaccination anti-covid pour toute la province Sud. Aujourd'hui, je suis inquiet. Très inquiet. Très inquiet. Quelques semaines après le deuxième référendum, le 4 octobre dernier, nous avons vu la Nouvelle-Calédonie s'embraser. Nous avons aussi assisté à des scènes proches de la guerre civile sur le dossier de rachat de l'usine Vale du Sud.

Mais je reste néanmoins préoccupé par ce qui peut arriver maintenant. Lors du deuxième référendum, le 4 octobre dernier, les bureaux de vote ont été pris d'assaut par des militants indépendantistes, drapeau identitaire kanak à la main, pour influencer, au pire pour dissuader, voire menacer, certains électeurs loyalistes. Il est clair, au vu de leur réaction pendant le conflit de l'usine du Sud, que les loyalistes ne vont plus subir en silence ces actions hostiles de la part de leurs adversaires. À quoi tout cela va-t-il nous mener ? Que se passera-t-il lorsqu'il y aura, devant les bureaux de vote, des militants de chaque camp qui considéreront qu'ils jouent là leur dernière cartouche ? Je pense que laisser se tenir un référendum binaire dans la situation actuelle, tel qu'il est prévu dans l'accord de Nouméa, alors que l'on sait que la population est divisée en deux et que l'on connaît le caractère explosif de la Nouvelle-Calédonie, c'est prendre un risque majeur pour l'avenir et figer de façon mortifère les oppositions ethniques, sociales et politiques. Monsieur le ministre, certains pourraient être tentés de simplement repousser la date du troisième référendum, au plus tard en septembre 2022, considérant que les prochains gouvernants traiteront ce sujet et que la Nouvelle-Calédonie ne représentera pas, dans ce cas, un risque majeur pour la campagne électorale. Ce serait une erreur Si le Gouvernement décidait de maintenir la même question que lors des deux premières consultations et de fixer la date au plus tard, la campagne présidentielle serait de fait instrumentalisée par les deux camps, et le moindre fait divers impliquant une ethnie contre l'autre serait utilisé pour servir sa cause. C'est un risque que vous ne pouvez pas faire prendre à notre pays et à la Nouvelle-Calédonie. Je porte, avec certains collègues, la conviction qu'une autre voie est possible. À plusieurs reprises, le pari de l'intelligence a été gagné en Nouvelle-Calédonie en 1988, au moment des accords de Matignon, où une entente improbable a été trouvée en quelques jours grâce à la volonté de Michel Rocard ; en 1998, en quelques semaines, parce que les responsables politiques locaux ont considéré que les plaies n'étaient pas suffisamment refermées pour organiser un nouveau référendum ; en mars dernier, au travers de l'accord sur l'usine du Sud, auquel plus personne ne croyait. autre voie, elle existe. Chacun en Nouvelle-Calédonie le sait. Indépendantistes et loyalistes savent que l'accord de Nouméa leur impose de se retrouver pour examiner la situation créée le lendemain du troisième référendum. Pourquoi attendre que les Calédoniens se déchirent une troisième fois pour rechercher cette solution ? Il est de la responsabilité du Gouvernement de poser un projet sur la table ; un projet qui maintiendra le lien si particulier que la France a construit depuis près de deux siècles avec la Nouvelle-Calédonie un projet qui reconnaîtra l'identité kanake et les autres identités qui cohabitent en Nouvelle-Calédonie ; un projet qui prendra en compte le fait que les divisions y sont à la fois géographiques, ethniques et politiques. Les accords de Matignon étaient fondés sur un partage du pouvoir entre les deux légitimités qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Ce partage géographique et politique a donné deux provinces sur trois aux indépendantistes et a permis dix ans de paix et de développement économique sans précédent. C'est lorsque l'accord de Nouméa a tenté de gommer les différences et de centraliser le pouvoir dans un gouvernement collégial que les choses se sont gâtées : dix-sept gouvernements en vingt-deux ans ! Sans commentaire

qu'il demande aux indépendantistes ce qu'ils attendent réellement de l'indépendance et aux loyalistes ce qu'ils veulent de la France. Le Gouvernement doit prendre le temps de rapprocher les solutions, avec la conviction qu'il ne peut pas échouer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très heureux que nous ayons ce débat, qui a été demandé par mon groupe. Il porte une double marque et veut adresser un double message. double message. Ce débat porte la marque de nos deux sénateurs calédoniens, même si je tiens à saluer tout particulièrement l'action de notre collègue Pierre Frogier et ses contributions. la marque du président du Sénat, dont chacun sait l'investissement personnel, au-delà de notre institution, à la résolution de la question calédonienne. Derrière l'attachement de Gérard Larcher, il y a aussi l'attachement jamais démenti de notre institution comme assemblée des territoires- territoire métropolitain, mais aussi territoires ultramarins.

Je ne conçois pas le destin de la Nouvelle-Calédonie comme étant différent du destin français. Le second message vous est adressé, monsieur le ministre, et, au-delà de votre personne, au Gouvernement. Dès lors que le processus des accords est en train de s'achever,

sociale, économique, mais aussi institutionnelle. Pour la première fois depuis plus de quarante ans, les mouvements indépendantistes se sont emparés de l'exécutif et ne parviennent pas à désigner un président pour le gouvernement. La crise institutionnelle

s'agissait. Nous qui refusons la partition entre la Nouvelle-Calédonie et la France, nous n'accepterons pas non plus de déplacer les frontières à l'intérieur du Caillou.

dangers un moment de tous les possibles et de tous les espoirs pour nous, mais surtout pour tous nos compatriotes néo-calédoniens, quelle que soit leur origine. La

dans la société civile intellectuelle, philosophique et spirituelle se sont mobilisés pour parvenir à ces accords. C'était quelque chose d'improbable, d'impossible presque,

vivant. Dans cette paix, au milieu de ces statues ancestrales, comment ne pas penser qu'il peut arriver dans l'histoire que le destin ne soit pas la haine, la guerre et la mort, mais que continuent de se lever contre les forces du mal

presse que des coutumiers bloquent une réunion politique du FLNKS, il faut méconnaître le dossier pour ne pas comprendre que la coutume et les coutumiers, autorité reconnue dans la République,

Certes, une initiative politique peut toujours émerger, mais jusqu'à preuve du contraire, le droit positif prévaut et parole a été donnée. Le premier référendum devait être organisé et il l'a été par le gouvernement d'Édouard Philippe.

une réponse de fermeté. Elle est là ! Moyennant quoi, il ne faudrait pas grand-chose pour que la justice et l'autorité judiciaire de notre République soient de nouveau regardées comme une « justice coloniale »- je cite ce que je peux lire dans les gazettes.

-de revenir sur cette distinction propre à nos institutions entre État et gouvernement. L'État est neutre ; le Gouvernement peut ne pas l'être.

Quelle est la définition de la pleine souveraineté ? Nous avons certes la définition que le droit international nous propose. Mais quand on discute avec les formations politiques indépendantistes,

ces sujets doivent être abordés avec patience et nécessitent beaucoup de temps. Vous avez tous noté que, si des accords ont été possibles en 1988 et en 1998, c'est parce que l'État était là. de ce que j'ai cru comprendre dans les propos des différents protagonistes, parce que nous avons su faire preuve à l'époque de tempérance, d'écoute, de dialogue et de compréhension à l'égard des aspirations les plus profondes des différentes parties.

Vous avez le dos large, monsieur le sénateur Frogier. Vous êtes expérimenté, et vous êtes un habitué de la vie politique calédonienne

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, malgré ses dégâts économiques et sociaux effroyables, la crise actuelle a pour mérite d'obliger les États et les entreprises à s'interroger sur l'organisation et la localisation de la production

pour le groupe auteur de la demande. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, malgré ses dégâts économiques et sociaux effroyables, la crise actuelle a pour mérite d'obliger les États et les entreprises à s'interroger sur l'organisation et la localisation de la production de biens et services présentant un caractère stratégique. L'épidémie de covid-19 nous oblige à questionner la logique de mondialisation. De fait, en délocalisant et en désindustrialisant, nous nous sommes privés de certains produits essentiels. Nous avons pris conscience de certaines illusions de la mondialisation heureuse. La pandémie a mis en lumière les risques inhérents à des chaînes de valeur fragmentées et mondialisées. Elle relance le débat sur le rôle de l'État, la nécessité d'une stratégie industrielle, et les risques économiques du « laisser-faire, laisser-aller ». Le sentiment de vulnérabilité du pays, qui a frappé nos concitoyens, a indéniablement ralenti l'élan, hier irrésistible, du train de la mondialisation. Reprendre en main notre destin commun ne veut bien sûr pas dire faire table rase du passé. D'ailleurs, les solidarités économiques construites ces quarante dernières années et nos engagements internationaux nous interdiraient de nous Cela implique toutefois de retrouver un État véritablement stratège, un État capable de définir les priorités essentielles et d'aider les entreprises à instaurer, là où c'est vital pour les intérêts stratégiques du pays, davantage de sécurité dans leurs circuits de production et d'approvisionnement. un État stratège plutôt que piètre gestionnaire ... Le Président de la République vient de se prêter au jeu consistant à imaginer la France de 2025. Il y évoque « l'excellence industrielle française, son nouveau modèle productif plus écologique et numérique ». Mais je m'étonne qu'il n'insiste pas sur l'urgente nécessité, d'une part, de garantir notre autonomie alimentaire et, d'autre part, de renforcer notre souveraineté dans le domaine de la sécurité sanitaire. Serait-il aveugle aux faiblesses de notre recherche, dont les ratés dans la mise au point d'un vaccin contre la covid-19 ne sont qu'un révélateur ? En janvier dernier, le Conseil d'analyse économique a examiné les raisons du retard français dans la course à l'innovation technologique, en mettant notamment en avant l'insuffisance des financements publics alloués à la recherche et à l'écosystème d'innovations. N'est-ce pas suicidaire à long terme ? Madame la ministre, comment comptez-vous rattraper ce retard ? Envisagez-vous, par exemple, de réduire la complexité du millefeuille administratif, le poids des normes et des procédures, de rapprocher les mondes de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée- tous ces thèmes que le Sénat défend depuis des années ? En bref, comment comptez-vous renforcer l'attractivité des métiers de la recherche ? Dans la high-tech et dans la biotech, les mêmes causes alimentent un retard français similaire. Ce n'est pas le moindre paradoxe de constater que les deux laboratoires parmi les plus en pointe, l'américain Moderna et le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, sont dirigés par des Français. Pourquoi a-t-on laissé partir Valneva au Royaume-Uni, alors que son siège était basé à Saint-Herblain et que cette entreprise de biotech franco-autrichienne va produire un nouveau vaccin ? L'été dernier, la start-up Snowflake a affolé Wall Street avec son introduction en Bourse record. Elle a été créée par deux ingénieurs français, qui ont trouvé leur bonheur au coeur de la Silicon Valley. Et n'oublions pas qu'Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de chimie en 2020, ne travaille plus en France depuis plus d'un quart de siècle. Elle y a pourtant été formée, a travaillé au sein des instituts Pasteur et Curie, des références mondiales dans ses spécialités. Et puis ... En tout cas, rien en France ! Pourquoi ne savons-nous pas suffisamment retenir nos chercheurs ou les faire revenir ? La maîtrise minimale de la souveraineté économique sous-entend que la prise de décision doit s'exercer au niveau de l'État-nation. Elle doit se conjuguer, bien entendu, en complémentarité avec nos partenaires membres de l'Union européenne. Si l'Europe peut être plus efficace dans certains domaines, alors appliquons-nous à développer une souveraineté européenne avec les partenaires prêts à nous rejoindre ! Sinon, vive le principe de subsidiarité Pionnières en matière de responsabilité sociale des entreprises, la France et l'Europe doivent se donner les moyens d'en défendre les principes et les règles. Il nous faut défendre les normes financières et extrafinancières- c'est-à-dire celles qui recouvrent des enjeux environnementaux, sociaux et de et de gouvernance -d'un capitalisme responsable. Réinvestissons dans le long terme ! Il y a aussi un préalable à la localisation ou la relocalisation d'activités en France améliorer les conditions de la compétitivité et de la productivité. C'est incontournable car, ne nous faisons pas d'illusion, la compétitivité par les prix reste le noyau dur des arbitrages, des individus comme des organisations. Cela vaut également, d'ailleurs, pour le prix des médicaments : la sécurité sociale est-elle prête à payer plus cher le paracétamol, par exemple ? Assurer la souveraineté économique, n'est-ce pas également préserver le tissu économique de la prédation d'entreprises étrangères ? Je pense aux nombreuses entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui sont ainsi menacées, alors même que la crise les fragilise. En trois mois, 500 d'entre elles ont fait l'objet de tentatives de prédation. Je pense aussi aux PME, nombreuses à être concernées par les 270 menaces identifiées par Bercy comme visant des entreprises de secteurs stratégiques au cours des dix premiers mois de 2020. Certains ont critiqué le refus de la France de voir le canadien Couche-Tard s'associer à Carrefour, ou encore l'interdiction du rachat de Photonis par l'américain Teledyne. Chacun peut avoir son idée sur les secteurs les plus stratégiques à surveiller. Pour ma part, je préfère que l'État soit vigilant sur ces sujets. Mais nous ne serons véritablement efficients que si nous arrivons à convaincre très rapidement nos partenaires européens de l'urgence à réviser les règles européennes de la concurrence. Celles-ci ne protègent pas suffisamment nos entreprises et les règles européennes des marchés publics ne les aident pas assez. En outre, le manque d'harmonisation fiscale et le niveau de la fiscalité française, y compris au moment de la transmission de l'entreprise, sont des obstacles supplémentaires. Quelles sont les priorités ? Comment les concrétiser et les financer ? Attention à la double injonction politique qui devient contradictoire dans certains territoires : relocalisation de l'activité industrielle et, « en même temps », application d'une politique « zéro artificialisation nette sans oublier d'autres entraves, comme la longueur des procédures d'urbanisme industriel ou commercial. Comment localiser ou relocaliser une entreprise, si l'on ne peut pas construire d'entrepôts Enfin, je voudrais insister sur un sujet majeur sur lequel la délégation sénatoriale aux entreprises travaille actuellement : la cybersécurité. Ce sujet nous concerne tous, individus, collectivités publiques, entreprises. Or ni la France ni même l'Europe ne sont souveraines dans ce domaine. Il n'existe même pas de européen souverain où stocker les données ! En France, 80 % des entreprises du CAC 40 et 75 % des entreprises du Next 40 sont clientes des services d'une multinationale américaine. Des entreprises stratégiques qui sont donc, par extension, soumises à la législation américaine du. Cette dernière offre un cadre légal à la saisie de documents, de mails et, plus largement, de toutes les communications captées à l'étranger par les serveurs des sociétés américaines. À quand un souverain, madame la ministre ? « Sans indépendance économique, il n'y a plus d'indépendance tout court », disait Charles de Gaulle ! La parole

portent sur les conséquences de la mondialisation et l'émergence de nouvelles superpuissances, que nous pensions, hier, simples ateliers du monde, ou d'entreprises numériques représentant des capitalisations pharaoniques. aussi sur les conséquences des choix stratégiques nationaux de ces trente dernières années, négligeant malheureusement des pans entiers de notre économie, notamment l'industrie.

pour s'étonner du déclassement de l'industrie pharmaceutique française en l'espace de deux décennies- cette dernière est passée de la première à la quatrième place et a perdu la moitié de sa part de marché mondiale -ou pour regretter des fermetures d'usines qui ont dévitalisé nos territoires. est venu, désormais, de travailler ensemble à la reconquête de notre souveraineté économique, et c'est tout le sens de la politique menée depuis le début du quinquennat par le Président de la République et la majorité présidentielle. L'impérieuse urgence de cette reconquête a été mise en exergue par la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Mais cette crise ne fait que révéler un état de fait, provoquant un effet de loupe sur des défaillances profondément ancrées dans notre pays depuis des décennies. Les difficultés d'approvisionnement en masques sanitaires, en médicaments, en matières premières stratégiques ou encore en intrants critiques essentiels, comme les semi-conducteurs, ont mis en lumière nos dépendances manifestes vis-à-vis d'autres continents. n'est pas uniquement français ; il est européen. La crise est le révélateur profond d'enjeux de souveraineté trop longtemps négligés. Soulignons que dans cette crise, et face à ces difficultés, nos industriels ont fait montre d'une formidable capacité d'adaptation, de souplesse, d'ingéniosité. Je tiens ici à les en remercier. Ils ont agi en lien étroit avec l'État et les collectivités locales, souvent en improvisant des partenariats inédits. Cela démontre la force de l'intelligence collective et du collectif, et c'est probablement sur ce type de modèles que nous devrions avancer. L'équilibre que j'évoquais précédemment doit aussi résider dans les solutions que nous avons à apporter, en nous méfiant des raccourcis et des amalgames. La souveraineté économique n'est pas le nationalisme mortifère ; la mondialisation et ses échanges sont, non pas des ennemis, mais des espaces dans lesquels nous devons inscrire notre action sans naïveté l'Europe n'est pas un handicap, bien au contraire, mais elle doit devenir notre principal atout et notre échelle de réflexion face aux puissances chinoise et américaine- pour ne citer qu'elles. Dès le début du quinquennat, sous l'impulsion du Président de la République, nous avons avec Bruno Le Maire engagé un mouvement de reconquête industrielle, d'investissement dans les compétences et les technologies de demain, de modernisation, de digitalisation de notre outil productif, pour que la France retrouve sa place parmi les grandes nations industrielles. Ce sont des premières mesures de refondation de notre économie qui ont été engagées, comme l'allégement de la fiscalité sur les investissements productifs, la suppression de cotisations sociales afin d'augmenter de façon directe, et non détournée, les salaires tout en baissant le coût du travail, la réforme des ordonnances Travail, qui facilite l'accès transformation des entreprises, dite Pacte, a renforcé le contrôle des investissements étrangers prédateurs pour protéger nos actifs stratégiques. Nous avons voulu rompre avec ce fatalisme qui consistait à faire de la France un pays d'économie post-industrielle, uniquement positionnée sur les services et qui jugeait notre industrie dépassée, polluante et incapable d'être compétitive. Nous voulons au contraire bâtir une industrie forte, innovante, décarbonée, participant à sa manière à la souveraineté des territoires et à leur continuité. Ces choix ont déjà permis de recréer des emplois industriels pour la première fois depuis 2000- en 2017, 2018, 2019 -et de redevenir le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers en matière industrielle en 2018 et 2019.

de la France, celle de l'Europe. Ainsi, 35 milliards d'euros seront destinés à soutenir notre industrie- nous faisons le pari de l'industrie ! J'ai bien noté que l'intitulé du débat n'évoque que la souveraineté économique française. Mais, à l'heure où les États-Unis et la Chine ont engagé des plans d'investissements massifs, je ne crois pas que nous rivaliserons seuls contre ces grandes puissances. La souveraineté française est indissociable de la souveraineté européenne. Nous avons besoin de plus d'Europe, mais surtout de « mieux d'Europe ». Il nous faut une Europe industrielle, ambitieuse en matière d'innovation, de transition écologique et de transformation des compétences, une Europe qui protège du dumping fiscal et environnemental, avec la mise en place d'une taxation sur les plateformes numériques, par exemple, ou d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une Europe qui impose une concurrence réellement loyale, à l'heure où des entreprises non européennes accèdent à des marchés domestiques sans contrepartie et sont fortement subventionnées.

Innover. Il s'agit là d'avoir le quart d'heure d'avance qui nous permettra d'être dans la cour des grandes nations industrielles en 2030, tout en nourrissant notre croissance actuelle.

vous avez évidemment mentionnée, s'inscrit dans un continuum avec l'innovation. Recherche fondamentale, recherche appliquée, tout l'enjeu de la loi de programmation de la recherche que nous venons de voter est

Cela doit aller de pair avec un cadre fiscal valorisant l'investissement productif. C'est le sens de la baisse des impôts de production, qui bénéficie, au premier chef, aux entreprises investissant sur les territoires.

aller de pair, enfin, avec un capitalisme français qui prend des risques. C'est le sens du fonds « French Tech Souveraineté » ou des fonds « Tibi », que nous orientons vers ces pépites industrielles. Mesdames, messieurs les sénateurs, nos territoires, que vous connaissez bien et que je sillonne quotidiennement, recèlent des atouts exceptionnels. Il nous appartient maintenant de bâtir une industrie puissante et une France en positif. C'est ce qu'attendent nos

Jean Bodin la définissait comme « le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint ». C'est une gageure au niveau économique. Loin de la volonté de tout faire soi-même et du mercantilisme, le Gouvernement a fait le choix d'une politique de souveraineté économique à la fois responsable et réaliste, avec ce qu'Emmanuel Combe et Sarah Guillou appellent dans une récente étude, d'une part, la « relocalisation des activités jugées stratégiques » et, d'autre part, une « politique industrielle de rattrapage technologique La stratégie pour le développement d'un hydrogène décarboné est un exemple concret de cette politique industrielle de rattrapage technologique. Lancée en septembre 2020, elle permet déjà à notre pays de se placer parmi les pays les plus en pointe dans cette technologie. Avec le soutien de France Relance- plan qui, rappelons-le, contient une enveloppe de 100 milliards d'euros -, les industriels et les territoires ont répondu à l'appel. Le 5 mars dernier, l'écosystème territorial hydrogène de l'Auxerrois, dans l'Yonne, a ainsi été présenté. Il s'appuie sur la création d'une station de production et de distribution multimodale d'hydrogène vert, issu exclusivement de sources renouvelables. La multiplication des hubs hydrogène dans nos territoires nous permettra de relever le défi de la souveraineté énergétique et industrielle, tout en décarbonant notre économie. Pouvez-vous, madame la ministre, nous apporter des précisions sur l'état d'avancement de la stratégie pour le développement de l'hydrogène décarboné ?

consommés en 2021 et 2022 afin de donner une impulsion à nos entreprises industrielles. L'enjeu est de créer les briques technologiques industrielles sur lesquelles on puisse s'appuyer pour, ensuite, déployer une véritable stratégie hydrogène dans deux directions

et accompagnera des consortiums réunissant des collectivités et des industriels fournisseurs de solutions pour favoriser au maximum des économies d'échelle, avec des projets ancrés sur les territoires.

d'une feuille de route stratégique européenne, qui concernera un certain nombre d'entreprises industrielles et nous permettra de gagner nos positions sur cette nouvelle technologie.

Le récent refus du rachat des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri ainsi que le refus du rachat du groupe Carrefour par un actionnaire canadien, s'ils sont bienvenus, ont montré une volonté de la part du Gouvernement de réaffirmer la souveraineté économique de la France. La crise de la covid-19 et les confinements qu'elle a engendrés ont encouragé de nombreux Français à revoir leur mode de consommation pour s'orienter vers des circuits plus courts et les acteurs locaux. Les scènes de rayons vides, la pénurie de masques au début de la pandémie ou encore les délais de vaccination, s'ils ne sont pas complètement imputables à notre stratégie économique, interrogent sur notre capacité à avoir un appareil productif performant pour répondre à la demande nationale. Ils interrogent d'autant plus qu'en parallèle la France est le pays européen ayant connu la plus forte désindustrialisation au cours des vingt dernières années, avec comme conséquences des délocalisations, de nombreuses suppressions d'emplois, l'automatisation et l'externalisation. Un seul objectif visé : réduire les coûts de production. Je parlais de concurrence mondiale, mais celle-ci est également européenne. Vous connaissez, madame la ministre, l'attachement de mon groupe à la construction européenne. Si la concurrence intraeuropéenne, qui est un fait établi, n'est pas près de s'arrêter au vu des différents coûts de production dans les États membres, seule l'Union européenne peut nous permettre de faire face aux géants que sont les États-Unis et la Chine. Aussi je vous poserai cette question : quelles solutions mettez-vous en oeuvre pour rendre possible la réindustrialisation et la souveraineté économique et alimentaire dans cette économie libérale mondialisée et dans une Europe concurrentielle ?

Au niveau européen, par ailleurs, on trouve tous les IPCEI- santé, souverain, hydrogène, microprocesseurs, batteries électriques -que nous avons lancés ou que nous souhaitons lancer dans les prochains mois. Nous

part, nous plaidons pour la coopération. Mais ne soyons ni les naïfs de la mondialisation libérale ni les Bisounours d'une Europe qui, non seulement se protège mal, mais organise en son sein une concurrence effrénée avec des dumpings sociaux et fiscaux. La France est particulièrement touchée. Il faudra bien changer ce cadre, mais, en attendant, il faut agir vite ! Si nous voulons inverser la spirale de désindustrialisation, de délocalisation, de détérioration grave de notre balance commerciale, en particulier avec nos partenaires européens,

Si nous avions eu des structures réellement opérationnelles, avec une mobilisation de tous les acteurs territoriaux et sociaux, avec une culture partagée partagée de l'intelligence économique, nous aurions certainement pu anticiper et éviter la vente d'une partie de notre fleuron national Alstom à General Electric et le démantèlement de Technip, qui passe sous pavillon américain.

Mais, plus inquiétant encore pour notre souveraineté économique, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions en matière de recherche. En effet, notre recherche scientifique est fondamentale pour notre souveraineté, car elle garantit notre capacité à innover. Notre indépendance passe par l'innovation, notamment dans la production pharmaceutique, comme j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler dans cet hémicycle en alertant sur nos vulnérabilités s'agissant des produits et équipements médicaux. La bataille économique se joue aujourd'hui sur le terrain scientifique et technologique. Une course s'est engagée et notre recherche nationale est notre meilleur atout pour favoriser les gains de productivité et la compétitivité. Toutefois, comme je l'évoquais, à l'automne dernier, dans mon rapport pour avis sur ce texte, la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a été une occasion partiellement manquée, ne donnant pas suffisamment à notre pays les moyens de rehausser son effort de recherche. Dès lors, madame la ministre, quel bilan faites-vous de cette loi ? Que proposez-vous afin que la recherche publique débouche sur la diffusion de connaissances nouvelles, notamment en lien avec la recherche privée, alors que la dernière loi de finances, certes en application de directives européennes, supprimait le doublement de l'assiette du crédit d'impôt recherche ? Quel rôle la recherche doit-elle jouer dans la bataille économique actuelle ? La parole

je tire de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche est plus favorable puisqu'est prévue une augmentation de 25 milliards d'euros des moyens destinés à la recherche sur les dix prochaines années.

et de nombre de fournisseurs étrangers pour des ressources hautement stratégiques- je pense notamment aux terres rares, si nécessaires aux industries qui font la compétitivité et donc les emplois d'aujourd'hui, et plus encore de demain -, quels sont selon vous les critères, les déterminants de la notion de souveraineté économique nationale ? Comment prenez-vous en compte la dimension européenne incontournable de ce concept ? On ne connaît bien, notamment pour y travailler, que ce que l'on mesure. Faute de quoi, on se paie de mots et on n'avance pas collectivement dans le bon sens, qui doit être celui d'un « confortement » de notre souveraineté économique nationale. Prenons un exemple,

Sa gouvernance, si elle est plutôt claire et rassurante pour la défense nationale, l'est beaucoup moins pour les acteurs économiques, les entreprises, grandes, moyennes et petites, dans notre territoire. Notre rapport l'a souligné et nous avons proposé que le Parlement discute, sur l'initiative du Gouvernement, une loi d'orientation et de suivi de la souveraineté numérique nationale.

à l'égard des producteurs asiatiques et chinois en particulier. La souveraineté économique de notre pays exige une stratégie industrielle et technologique à long terme. La France dispose d'atouts pour relever ce défi. Certes, elle peut et elle doit s'appuyer sur ces filières d'excellence. Les dynamiques d'innovation des entreprises françaises sont les premiers supports de cette ambition. Notre pays doit aussi mobiliser les leviers européens pour renforcer sa souveraineté économique et industrielle. L'an dernier, j'ai été interpellé par une entreprise de taille moyenne, qui avait le projet d'implanter une usine de production d'hydrogène par électrolyse d'eau. Elle ambitionnait d'intégrer un projet IPCEI, véhicule précieux qui autorise des synergies européennes dans un cadre assoupli en matière d'aides d'État. Seul un soutien public pouvait permettre de développer cette initiative qui devait conduire à la création d'emplois locaux. La France doit appuyer la création de ces outils européens et faciliter leur mise à disposition pour faire émerger des leaders industriels dans des filières innovantes comme celles de la production d'hydrogène ou des semi-conducteurs. Les acteurs industriels sont prêts à s'en saisir et les collectivités souhaitent s'y associer pour le développement économique de leurs territoires. La France doit aussi s'atteler à obtenir un soutien financier de l'Europe, bien sûr, pour ces filières d'importance stratégique. La négociation en cours de la taxonomie verte est à cet égard décisive. Il s'agit de définir le périmètre des investissements nécessaires à l'accompagnement de la transition climatique. Si la filière nucléaire en était exclue, c'est tout l'avenir de cette filière d'excellence française qui se trouverait compromis. C'est un enjeu essentiel d'autonomie stratégique. Madame la ministre, comment le Gouvernement entend-il faire de notre appartenance à l'Union européenne un levier pour la compétitivité de notre industrie, pour l'emploi et la vitalité de nos territoires et, finalement, pour la souveraineté économique de la France ?

prochaines semaines. Mais nous devons l'accompagner d'autres projets. C'est pourquoi nous portons des projets en matière de santé, de souverain,

Tout en saluant la pertinence et la nécessité d'un tel débat, je souhaite rappeler que cette souveraineté peut bien être envisagée au niveau national mais également, et surtout, au niveau européen. Comme dans les autres domaines, la France doit assurer sa souveraineté en matière économique. Travailler avec nos partenaires européens nous permettra de développer des solutions efficaces et pérennes. Notre dépendance dans le domaine industriel a été mise en lumière au plus fort de cette crise sanitaire. Au cours des dernières années, nous avons laissé beaucoup de filières s'affaiblir, quitter notre territoire. La France est donc l'un des pays les plus touchés par Ces délocalisations se sont traduites par une dépendance accrue de notre pays dans plusieurs domaines. Nous sommes nombreux à souhaiter qu'il retrouve le contrôle de ses capacités de production. Notre industrie doit cependant faire face à une concurrence déloyale, notamment en matière écologique. À cet égard, la filière sidérurgique me semble emblématique : la part de l'acier européen n'a cessé de reculer dans la production mondiale, rendant l'Europe de plus en plus dépendante en la matière. Les concurrents de notre industrie ne sont pas tous astreints aux mêmes obligations de réduction de gaz à effet de serre. En mars dernier, le Parlement européen a voté le principe d'une taxe carbone aux frontières pesant sur les importations. Cette taxe doit permettre de concilier la poursuite des objectifs de préservation de l'environnement et de localisation de la production européenne.

d'acier en provenance de pays qui n'ont pas les mêmes modèles sociaux et environnementaux que les nôtres. Leurs entreprises, de surcroît, ont pu bénéficier d'une certaine forme de soutien, soit par un accès privilégié au marché domestique-

C'est tout particulièrement le cas concernant la gestion des déchets. Création d'emplois, savoir-faire des salariés, circuits courts, recyclage, respect de l'environnement, écologie de pointe : avec tous ces atouts pour l'économie française, ce secteur d'avenir est malgré tout, depuis plusieurs années, en danger.

Depuis février 2020, les salariés ont lutté pour le maintien du site. Alors que celui-ci aurait pu être converti en bijou écologique grâce à l'expertise des salariés, il y a eu plus de 250 licenciements en juillet dernier, et le site risque d'être démantelé dans huit semaines. Il est donc temps de passer de la parole aux actes. Le Gouvernement doit soutenir les salariés, qui souhaitent changer les habitudes des modes de production, tendre vers une industrie écologique et radicale créatrice d'emplois, qui rompt avec la logique passéiste dont on connaît trop bien les ravages à la fois sociaux, climatiques et environnementaux. UPM reste propriétaire de cette usine, l'État doit favoriser les dossiers qui promeuvent la papeterie écologique et le recyclage des déchets. Il faut une réponse sur un sujet global : la collecte des filières de recyclage. Alors que le plan de relance prévoit 30 milliards d'euros pour la transition écologique et que le ministre Bruno Le Maire annonçait, l'année passée, que cette dernière devait être l'horizon de notre économie, le Gouvernement ne donne aucune réponse sur l'avenir de la filière du papier recyclé en France et, plus largement, sur les projets industriels tournés vers les sujets environnementaux. Nous regrettons ainsi l'absence totale de contreparties sociales et environnementales pour notre économie. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que la papeterie Chapelle Darblay, fleuron de l'économie circulaire, demeurera un site spécialisé dans le secteur de la gestion et du recyclage des déchets réels

Darblay, dont vous avez raison de dire qu'il coche toutes les cases en matière de transition écologique et d'industrie. Le Gouvernement s'est engagé à lever les obstacles à la reprise et à accompagner le projet dans le cadre du plan de relance. Pas plus tard que le 30 mars dernier, j'ai pris des engagements écrits en en signant un courrier de confort à deux repreneurs potentiels, leur assurant qu'une partie des investissements nécessaires à la reconversion de l'usine Chapelle Darblay devraient être financés sur les crédits du plan de relance.

pour que, le 15 mai, les projets de reprise soient définitifs, afin de donner un avenir aux salariés et au territoire. Nous travaillons main dans la main avec les organisations représentatives du personnel et les élus locaux.

confiées toujours et encore à l'américain Palantir. Je pense enfin aux prêts garantis par l'État (PGE), confiés à Amazon Website, qui dispose donc aujourd'hui d'informations stratégiques sur les entreprises françaises et peut ainsi cibler les acquisitions opportunes pour des investisseurs étrangers hors Union européenne. Ces géants américains du numérique, nous le savons, ont un savoir-faire technologique indéniable. Amazon investit chaque année 22 milliards d'euros dans la recherche et le développement. Mais nul besoin, madame la ministre, de rappeler les dispositions extraterritoriales du en matière de transfert des données aux États-Unis. Nul besoin non plus de rappeler qu'Amazon Website gère le de la CIA et de l'organisme américain chargé de la régulation et du contrôle des marchés financiers. Si nous voulons réellement, au-delà des mots, reconquérir notre souveraineté numérique et donc économique, l'achat public doit devenir le levier majeur de la politique industrielle française, y compris pour le numérique, comme les États-Unis le pratiquent eux-mêmes depuis des années avec le succès que l'on connaît. L'État ne doit-il donc pas, madame la ministre, soutenir et privilégier davantage les offres souveraines existantes et équivalentes ou presque à l'offre américaine et dépasser cette forme de défiance que nous avons à l'égard de nos propres acteurs français de l'écosystème et que l'on observe malheureusement depuis un certain nombre d'années Quelle place également pour le européen Gaïa-X, tant attendu, qui se révèle être davantage une base de données et de logiciels unifiée dans le but de les connecter qu'un outil de souveraineté numérique européenne destiné à protéger les données des Européens ? La parole est à Mme la ministre

et aux sociétés politiques qu'il appartient d'y mettre de l'ordre et de la justice : notre débat de ce jour sur la souveraineté économique de la France nous renvoie à cette évidence. Cela étant, pour être

est majeure aujourd'hui. Il est donc essentiel de faire émerger, en Europe, de nouveaux acteurs du numérique dont les activités respecteraient les principes et les valeurs des Européens. Aujourd'hui, le développement de l'industrie numérique et digitale impose sans doute une mise en ordre de l'effort national, mais dans une logique de coopération ouverte et européenne. il convient de constituer le cadre réglementaire pour circonscrire l'activité des entreprises et des professionnels de ce secteur. Il est également nécessaire de garantir les droits et libertés de nos concitoyens et la capacité d'action des autorités publiques de régulation. D'un point de vue industriel, comment l'Union européenne et la France contribuent-elles à créer un écosystème vertueux susceptible de constituer demain une concurrence européenne aux Gafam et aux BATX vous l'entendre dire, se résigner à ce que la bataille soit définitivement perdue ? Plus précisément, où en est la mise en oeuvre de l'initiative européenne sur l'informatique en nuage, l'acquisition de calculateurs à haute performance de nouvelle génération et le développement de la technologie quantique ?

soutenir le développement de l'offre de la filière industrielle du et promouvoir l'interopérabilité ; soutenir la recherche, le développement et l'innovation dans les domaines du présentant un fort potentiel de création de valeur, comme l'intelligence artificielle,

3 000 entreprises. Accessoirement, il produit 70 % de notre électricité ... Las, les petits arrangements politiques et le manque de décisions anticipatrices

Au coeur de l'été 2019, il annonçait même l'arrêt du programme Astrid, dédié aux réacteurs de quatrième génération. Sur ce dernier point, je mène depuis plusieurs mois une mission pour l'Office Sans dévoiler les conclusions de ce travail, je tiens à déplorer le coup de frein brutal infligé à la recherche nucléaire. En la matière, la France était le leader incontesté depuis de nombreuses années ; mais, aujourd'hui, elle ne représente plus une hypothèse incontournable pour nombre de projets internationaux.

dans le dispositif d'appel à projet Résilience, qui vise à permettre des relocalisations industrielles en France. J'en veux également pour preuve les 470 millions d'euros que le plan de relance

qu'EDF va abonder à hauteur de 100 millions d'euros, et un programme de renforcement et de modernisation des compétences des appels à projet et des manifestations d'intérêt. L'enjeu est de former

M. le ministre Bruno Le Maire déclarait il y a peu que « la France entendait se montrer très vigilante quant à ces projets de rachats qui menacent la souveraineté européenne permettez-moi de vous donner un exemple qui illustrera parfaitement mon propos et l'objet du débat de ce jour. L'entreprise ariégeoise Aluminium Sabart, fleuron de l'industrie française pour la production d'aluminium de haute qualité,

Pourtant, très rapidement, les inquiétudes ont resurgi : le groupe chinois semble faire table rase de ses belles promesses. En effet, après la fermeture du site d'Alfisa, le placement en redressement judiciaire de la SAM et de la FVM,

À ce titre, quelles sont les armes, tant d'anticipation que de contrôle, dont dispose l'État pour défendre les actifs stratégiques nationaux ? La parole

pour nous, est de trouver une solution industrielle pour ce site. Vous avez raison de mentionner la situation dans laquelle se trouve la fonderie SAM, elle aussi reprise par Jinjiang à la barre du tribunal.

Je ne peux que me réjouir de la tenue de ce débat, alors même que la souveraineté économique était, il y a encore peu, le pire des blasphèmes. La souveraineté économique, c'est la capacité d'un État à maîtriser son destin économique en assurant son indépendance dans des secteurs stratégiques. C'est aussi une certaine idée de la protection des Français. Pourtant, l'industrie du médicament, secteur éminemment stratégique, se porte mal en France. Il faut se le dire : notre pays n'est plus souverain en la matière l'excellent rapport de notre collègue Jean-Pierre Decool mettait en lumière les pénuries de médicaments et de vaccins. La crise sanitaire n'a fait que confirmer les conclusions de ce travail. Qu'il s'agisse de traitements lourds et durables ou de médicaments aussi quotidiens que le paracétamol, la France souffre régulièrement de pénuries. À de multiples reprises, j'ai attiré l'attention du Gouvernement sur ce problème, en prenant comme exemple le cas d'UPSA, lot-et-garonnais qui continue à souffrir d'une politique déraisonnable du prix du médicament. Pourtant, cet acteur de premier plan a su se mettre au service de la France pour faire face à la pénurie de paracétamol.

d'euros. Madame la ministre, qu'en est-il de vos promesses ? Où en est le plan présenté le 18 juin 2020, visant à rapatrier les industries de santé stratégiques sur le territoire national dans les trois ans ?

actes, car une promesse c'est comme une fonction : il faut l'honorer quoi qu'il en coûte

La France importe encore à ce jour 20 % de son alimentation, dont 25 % de la viande de porc, 34 % de la volaille, 50 % des protéines végétales et des fruits. Si nous n'avons fort heureusement pas souffert de pénuries du fait de la crise sanitaire,

L'immense majorité de ce budget vise à augmenter les capacités de production agricoles. Il serait pourtant naïf de penser que ces crédits suffiront pour restaurer la souveraineté économique de la France en matière d'agriculture. Un ensemble de facteurs doit être pris en compte et les investissements ne doivent pas tous être fléchés vers des machines permettant de meilleurs rendements ou l'augmentation des surfaces agricoles. Le terrible épisode de gel que nous avons connu il y a quelques semaines en est d'ailleurs le parfait exemple sans investissement dans la résilience de l'agriculture face au changement climatique, l'augmentation de la production est réduite à néant. De même, sans éducation de la population- il faut expliquer pourquoi les prix de l'agriculture française peuvent être plus élevés tout en insistant sur les bienfaits d'une consommation locale -, nos efforts sont vains.

Madame la ministre, comment prévoit-on d'aider l'agriculture à s'adapter au changement climatique ? Comment comptez-vous inciter à la consommation française ? Allez-vous investir plus massivement dans la recherche pour que la souveraineté alimentaire française ne reste pas une pure utopie ? La parole est à Mme la ministre

Résilience ! La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier. Plus que jamais, la révolution du représente un péril pour la souveraineté de la France. Tous les jours, les Gafam se livrent à un véritable pillage en exploitant massivement les données de millions de Français. Soumis à des lois extraterritoriales, ces géants du numérique sont désormais des entreprises systémiques, capables de concurrencer les États. Comme l'expliquait déjà notre collègue Gérard Longuet dans son rapport d'octobre 2019, les Gafam menacent le monopole fiscal de la France. Avec une capitalisation boursière qui correspond à plus de deux fois celle du CAC 40, le chiffre d'affaires des Gafam est désormais comparable aux recettes fiscales françaises. Réponse nécessaire, mais insuffisante, du Gouvernement, la taxe sur les services numériques instaurée en 2019 n'a répondu que partiellement au défi fiscal posé par les entreprises du numérique. Ces dernières continuent d'échapper largement à l'impôt.

étant, la lutte pour la souveraineté numérique de la France ne se résume pas à l'harmonisation interétatique de la taxation des Gafam. Reprendre le contrôle de notre souveraineté numérique suppose aussi d'organiser le rapatriement des données de nos concitoyens et des entreprises françaises sur le territoire national. Aujourd'hui, 92 % des données occidentales sont hébergées aux États-Unis. Afin de garantir la sécurité économique de nos entreprises, il est primordial de sortir de cette situation de dépendance numérique en proposant des solutions d'hébergement sûres, réparties équitablement sur l'ensemble du territoire national. Enfin, la France doit impérativement capitaliser sur l'expertise de ses ingénieurs en développant un modèle économique compétitif fondé sur les technologies digitales de pointe. C'est à cette unique condition que notre pays pourra sortir de sa position de colonisé numérique et créer des gisements de croissance grâce au levier du digital. au levier du digital. Quel plan le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour pallier le désarmement numérique de la France et atteindre l'indépendance technologique dont dépendent la sécurité et la souveraineté économiques de ses entreprises

souverain européen ! La parole est à M. Bernard Fournier. Malheureusement, comme souvent, il aura fallu une crise historique pour que, collectivement, nous nous rendions compte à quel point notre pays était devenu dépendant sanitairement, industriellement et, au total, économiquement d'autres grandes puissances. Que n'ai-je pas entendu ces dernières années, ici même, dans cette assemblée, quand nous parlions de la désindustrialisation de nos territoires, de la défense de notre souveraineté, de la protection de nos entreprises, qui se faisaient racheter une par une ; quand nous défendions la branche énergie d'Alstom, (ADP) ou encore Photonis, dont personne ne parlait ? Nous étions des conservateurs, des souverainistes qui n'avaient rien compris à la mondialisation, au commerce international ou aux règles du libre-échange Aujourd'hui, je souhaite tout simplement pour notre pays, et plus largement pour l'Europe, que nous fassions preuve de plus de réalisme et de pragmatisme. Les Français, légitimement, comprennent de moins en moins notre naïveté face à des pays comme la Chine ou les États-Unis, qui utilisent toutes les armes économiques, douanières, fiscales ou monétaires pour se protéger et qui investissent massivement chez nous. Nous pouvons le regretter, mais, depuis plusieurs années, tous les grands pays se referment et renforcent leur législation pour mieux protéger leurs entreprises des rachats par des investisseurs étrangers. En France, depuis 2014, nous avons élargi le décret qui soumet certains investissements étrangers à l'autorisation du Gouvernement. Ces mesures, que vous avez encore améliorées, madame la ministre déléguée, ne suffisent pas, car nos groupes sont particulièrement vulnérables depuis la crise du covid. Nous devons trouver un chemin étroit et difficile entre la protection de nos entreprises et une économie ouverte, attractive, dans plus de 2 millions d'emplois dépendent de groupes étrangers installés sur notre territoire. Aussi, je souhaiterais que vous nous précisiez la politique que met en oeuvre le Gouvernement pour que la France protège plus efficacement ses entreprises, notamment

a aussi inspiré la doctrine de filtration des investissements en Europe, dont on peut penser qu'elle pourrait aller plus loin, mais qui, à tout le moins, nous permet d'échanger des données, comme nous avons pu le faire avec l'Italie, sur le dossier Iveco.

de General Electric, Bruno Le Maire a annoncé travailler à une solution souveraine sur la partie Arabelle Liberty, c'est précisément parce que les conditions relatives aux investissements étrangers en France sont très fortes que nous avons pu obtenir un certain nombre de mouvements et préserver

suivi 275 opérations de contrôle sur les IEF, ce qui montre l'efficacité du dispositif, et nous sommes prêts à aller plus loin.

C'est le cas de l'impératif de souveraineté économique. Après des décennies de mondialisation, l'indépendance économique totale est un objectif qui ne peut être atteint, et qui n'est pas même souhaitable. Les liens économiques qui nous unissent à nos partenaires sont denses, innombrables, bénéfiques pour notre économie, sources d'innovation, de conquête, d'ouverture et sont donc inaltérables. La question centrale, celle de la souveraineté, reste néanmoins valable est-elle en mesure, aujourd'hui, d'assurer ses propres besoins fondamentaux, ceux de l'État et ceux de ses citoyens, quels que soient les risques géopolitiques, commerciaux ou, on l'a vu, sanitaires ?

reposent sur un équilibre fragile que les tensions géopolitiques et commerciales peuvent faire vaciller. Or nous savons- car c'est là une politique assumée -que des pays comme la Chine, mais aussi les États-Unis, regardent avec intérêt nos meilleures entreprises et nos savoir-faire uniques. Je vous ai alerté sur ce point, alors que vous insistiez pour faire aboutir la vente des Chantiers de l'Atlantique à Fincantieri, associé à l'entreprise d'État chinoise CSSC. Que dire de la vente d'Alstom à General Electric ? Une fois ces transferts de technologie réalisés, que nous restera-t-il ? Nous résumons souvent la souveraineté économique à la sauvegarde des biens et des services nécessaires à nos activités régaliennes : à la défense, aux communications,

est celle d'hier ; il nous faut voir plus loin. La souveraineté économique n'est-elle pas aussi la défense de notre potentiel économique national, de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos start-up, de notre tissu productif,

Je me permets de vous suggérer d'associer les territoires à votre réflexion. Ceux-ci savent identifier leurs besoins et leurs atouts, on l'a vu durant la crise. La qualité d'un tissu économique tient aussi à l'infrastructure, à la formation et aux services publics : les collectivités jouent là un rôle de premier plan. Des entreprises structurantes sur le plan local peuvent être des piliers de la souveraineté économique ; un capitalisme territorial rénové peut être un levier fort. Enfin, il nous faut protéger juridiquement nos entreprises face à la législation de face à la législation de pays puissants usant de l'extraterritorialité de leur droit, décidée unilatéralement. Nos amis américains ou chinois sont redoutables ; ils sont nos amis,